Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué il y a pas d'observation, le procès verbal est adopté sous les réserves d'usage. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture est parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales et la parole est à monsieur Stéphane Sautarel. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, la ministre ma question pardon été adressée à la ministre chargée des collectivités rurales et de la ruralité. Je souhaite en effet attirer votre attention sur la situation des syndicats de communes concernées par le transfert de la compétence eau et assainissement. Qui soit existants et surtout à créer la loi notre de 2015, modifiée en 2018 a prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération au 1er janvier 2026, l'article 14 de la loi de 2019 relatives à l'engagement de proximité autorise les communautés de communes. Ah déléguée par convention tout ou partie de ses compétences à une commune ou à un syndicat infra-communautaire existant au 1er janvier 2019, qui ont fait la demande. La loi 3DS quant à elle, voté il y a un an renverse ce principe en prévoyant que pour les communautés de communes qui deviennent compétentes à titre obligatoire au 1er janvier 2026 les syndicats infra-communautaire ayant ces compétences soient désormais maintenu par la voix de la délégation, sauf si les communautés de commune délibère contres se maintient. Ainsi, faute de garantir la liberté locale du mode de gestion aux communes de nos territoires que j'espère nous pourrons encore établir d'ici 2025. Il convient d'éviter le risque d'un mitage obligeant Obligeant les EPCI soit à refuser toute délégation soit à à naître un acteur partiel ce qui sera déjà le cas d'ailleurs avec les syndicats. Terre départementaux alors que de nouveaux syndicats intercommunaux souhaite se mettre en place de manière concertée il importe qu'il puisse le faire voir y être incité pour que leur soit déléguer les compétences eau et assainissement. Je vous remercie donc de préciser les modalités pratiques et les délégués et les délais qui serait prévu par voie réglementaire à cet effet et les instructions données aux préfets pour ses créations postérieure au 1er janvier 2019. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Stéphane. Sautarel. Vous le savez, la montée en puissance de l'intercommunalité sur la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise en perspective du dérèglement climatique et des enjeux de la gestion de l'eau et des enjeux de la gestion de l'eau potable car elle vise à exercer cette compétence à un échelon de mutualisation et de solidarité. La loi du 27 décembre 2019, dite loi engagement et proximité autorise ainsi les communautés de communes et communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau Au 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS ces syndicats infra-communautaires seront maintenus par voie de délégations sauf vous l'avez rappelé délibération contraire de la communauté de communes. Il est important de noter que dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence délégué qui est exercée à son nom et pour son compte. La communauté de communes et donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, qu'elle soit ou non délégué en partie à un syndicat infra-communautaire. Existant au 1er janvier 2019. S'agissant de la création d'un syndicat exerçant ses compétences après le 1er janvier 2019. Rien ne l'interdit. Dès lors que 2 conditions sont respectées. Que sa création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale. Et qu'il s'agisse d'un syndicat dont les limites territoriales dépasse le seul périmètre de la communauté de communes, il ne peut s'agir d'un syndicat. Infra-communautaire. Dans le cadre de la création d'un tel syndicats la communauté de communes et substituer pour les compétences qu'elles exercent aux communes qui en sont membres. Je vous remercie. Non il y a que 4 secondes alors. C'est pas possible. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier. Merci Merci madame la présidente, monsieur le ministre du logement. Je souhaite vous interroger sur la politique de construction de logements sociaux dans les territoires ruraux. En effet, de forts besoins en logements sociaux existent dans les territoires. Ces logements permettent d'accueillir une population vieillissante mais également des familles familles monoparentales, des jeunes actifs. Pourtant de nombreuses difficultés viennent ralentir, voire stopper les projets de logements sociaux dans nos communes rurales en effet l'inflation et l'augmentation du coût des matières premières pour la réalisation des travaux, un impact Direct sur des projets pour la plupart déjà plus coûteux qu'en zone urbaine. Les bailleurs sociaux sont également impactées par l'augmentation du taux du Livret A qui est passé de 0,5% à 3% en un an, ce qui alourdit les charges d'intérêt des organismes de logement social de 3,75 milliards. Enfin la réduction du loyer de solidarité mis en place en 2018 pour compenser la baisse des aides au logement. Et qui grèvent les Budgets des bailleurs a un impact plus fort en milieu rural. Cette situation a pour conséquence d'entraîner le désengagement de bailleurs sociaux. Vous donne l'exemple de la commune d'appuyer dans mon département de la Mayenne, une commune. D'un peu moins de 1000 habitants. Qui connaît une croissance démographique dynamique. Elle avait un projet de 4 logements sociaux avec un permis délivré, il y a plus d'un an. L'appel d'offres du bailleur social arrive à une augmentation avec un coût prévisionnel à plus 12% nécessitant une mobilisation des fonds propres 3 fois supérieur à ce qui est consenti habituellement la conséquence c'est l'ajournement du projet. Pour autant, les besoins en logements. Sur la commune sont sont toujours présents, une forte attente logement social mais pas seulement. Parce que nous on a un besoin pour pour les habitants. Moins d'habitants, c'est aussi une problématique pour nos écoles rurales qui font face dans l'État à des fermetures de classes. Donc Monsieur le Ministre, quelle position qu'est le soutien du gouvernement pour la construction de logements sociaux dans ces communes rurales qui n'ont pas les moyens de les financer. Merci. La parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Guillaume Chevrollier. Vous le savez, les bailleurs sociaux sont d'ores et déjà présent fort heureusement en zone rurale. Au cours de l'année 2022, il y a eu plus de 16.203 logements locatifs sociaux en offre nouvelle agréé en zone rurale. Pour faire face à la hausse du coût des travaux que vous soulignez les montants moyens de subvention par logement locatif en offrent nouvelles ont été revalorisée de 5,4%, à l'échelle nationale pour l'année 2023. Cette revalorisation est modulée entre les régions et à l'échelle infra-. Par ailleurs, le gouvernement continue à promouvoir l'acquisition amélioration et en particulier dans les territoires détendu qui concerne 74% du parc privé durablement vacants. L'acquisition amélioration et représente un levier important pour créer une offre nouvelle de logements locatifs sociaux cohérente avec les objectifs de diminution de l'artifice la deux l'artificialisation. Des espaces agricoles naturels et forestiers et qui participent à la dynamisation de nos territoires. Pour cela une dotation de 23 millions d'euros dédiée aux opérations d'acquisition amélioration difficile à équilibrer financièrement a été créé en 2022. En 2023, cette dotation est élargie à toutes les opérations participant à à la sobriété foncière de l'offre nouvelle de logements locatifs sociaux et son montant a été relevé à 45 millions d'euros. La revue utilisation des centre-ville centre-bourg fait l'objet d'un fort soutien du gouvernement, notamment dans le cadre des programmes Action coeur de villes dans lesquelles la réhabilitation des logements peut bénéficier d'aides importantes. Enfin la lutte contre la vacance des logements en milieu rural et l'amélioration du parc devrait être des axes clés du second souffle de l'agenda rural en cours d'élaboration. Je vous remercie. Merci alors. La parole est à Madame Dominique Estrosi Sassone. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la délégation aux communes de la compétence zone d'activité économique. Si la loi 3DS apporte un certain nombre d'assouplissement pour les transferts de compétence la compétence concernant les zones d'activités économiques n'a pour l'heure fait l'objet d'aucune modification depuis la loi de notre cette compétence est obligatoirement transférée aux EPCI à fiscalité propre. Pourtant il existe des cas de figure pour lesquels le transfert permettrait aux communes de porter des projets plus efficacement que le PCI. Je prends à dessein l'exemple de la commune de toiture var dans mon département qui est propriétaire d'un terrain classé zone d'activité au PLU et cela, en parfaite cohérence avec le Scott de la communauté de communes des Alpes d'Azur. La commune souhaite y réaliser une zone artisanale. Le maire a d'ores et déjà obtenu une subvention de l'État et de la région. Mais lorsqu'il a été question de la taxe sur la valeur ajoutée puisque les opérations d'aménagement comportant des cessions de terrains sont assujettis de plein droit à la TVA. Il a été précisé au maire que cela a été impossible puisque la compétence relever de l'EPCI. Or, la communauté de communes en question ne dispose pas des fonds pour réaliser cette zone artisanale et le terrain il appartient lui toujours à la commune ainsi que les subventions obtenues sont bien au nom de la commune. Monsieur le Ministre, entendez-vous revoir la législation afin que le transfert de compétences soit possible dans le cas d'une commune volontaire ou a minima permettent d'autoriser une possibilité de sub-, délégation de l'EPCI à la commune en vue d'obtenir une autorisation pour réaliser certains aménagements comme une zone d'activité économique. la parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente. Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice. Dominique Estrosi Sassone vous l'avez rappelé depuis la la loi notre les. PCI à fiscalité propre exerce sa compétence obligatoire de création d'aménagement d'entretien et de gestion des zones d'activités économiques en effet. Ils sont identifiés comme l'échelon le plus à même de créer et de gérer des zones d'activités à l'échelle pertinente du bassin de vie économique pour un développement équilibré du territoire. La loi 3DS du 21 février 2022 que vous citez permet à un EPCI à fiscalité propre avec l'accord de ses membres de déléguer à un département ou une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transféré cette possibilité qu'on cerne les compétences facultatives. Vous le comprendrez. Et la position du gouvernement et constante sur ce point, il n'est pas envisagé de revenir sur l'attribution de la compétence de développement économique au niveau intercommunal. Cet acquis de la loi notre permet de porter des projets plus ambitieux et de rationaliser la création de zones d'activités à l'échelle de territoire plus vaste de nombreux outils existent toutefois pour assurer une meilleure association des maires à la décision au sein de leurs EPCI à fiscalité propre. La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 a par exemple permis l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les et PCI et les communes membres. Ce qui peut favoriser une meilleure concertation en amont sur ce type de projet. Le dialogue entre la commune et son EPCI concernés devraient permettre de statuer sur l'avenir de ce projet ou d'en organiser la reprise par le PC. Je vous remercie. Merci madame Estrosi Sassone vous avez 9 secondes. Oui j'entends tout à fait des arguments de Monsieur le Ministre, je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour mais je pense qu'il faudrait voir ça plus dans le, dans le détail parce qu'en l'occurrence ici, il s'agit d'une communauté de communes qui est de taille assez modeste et avec des communes qui elles ont la possibilité de réaliser ces zones d'activités artisanales et pas une communauté de communes. Donc je pense vraiment. Merck qu'un assouplissement ferait du bien à certains. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Pierre Louÿs. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de la Transition écologique. En avril 2020, le gouvernement a souhaité limiter les facteurs de transmission du Covid en imposant un traitement hygiénique supplémentaires avant d'épandage agricole des boues de stations d'épuration. Des collectivités publiques ont alors massivement investi pour moderniser leurs stations et notamment grâce à l'aide d'une subvention exceptionnelle de l'État. Soulignons qu'elles subissent. Par ailleurs, la pression de l'augmentation du prix de l'énergie et du point d'indice des fonctionnaires mais aujourd'hui et ne perçoivent plus d'aucune subvention de l'État. De plus, au cours d'un rapport publié en octobre 2022, le Conseil de la santé publique a conclu qu'il ne semblait pas nécessaire de maintenir des mesures restrictives d'épandage des boues actuellement en vigueur. J'ai appris ces derniers jours que la signature pour l'arrêt de ses traitements était imminente. Je souhaiterais donc savoir si vous confirmez bien l'abrogation des arrêtés du 30 avril 2020 et 20 avril 2021. aux restrictions d'épandage des boues. C'était une application disproportionnée du principe de précaution qui aura coûté plusieurs millions d'euros aux collectivités locales. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Pierre lourd. Du fait du risque de propagation du virus lors de l'épidémie de Covid 2019 les conditions d'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles ont été effectivement modifié pour prévoir une hygiène Isa Sion ou un traitement des boues avant leur épandage pour aider les collectivités compétentes en matière d'assainissement à supporter les dépenses liées à ces nouvelles conditions d'épandage. L'État a rapidement mis en place un dispositif de soutien financier exceptionnel par l'intermédiaire des agences de l'eau. Pour les années 2021 et 2022, les investissements nécessaires à la gestion des boues ont ainsi été pris en charge dans le cadre du plan de relance, ce qui a par ailleurs été sans incidence sur la capacité des agences à accompagner financièrement les collectivités dans leur projet d'assainissement. En juillet 2022, compte tenu de l'évolution favorable de l'épidémie, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a ainsi saisi le Haut Conseil de la santé publique afin de savoir si ces mesures pouvaient être désormais amoindris voire totalement levé. Dans son avis du 21 octobre 2022 le H. S. C.. Sp s'est montré favorable à la levée des restrictions en matière d'épandage des boues. En période de Covid, telle que fixée par l'arrêté du 30 avril 2020 modifié le 20 avril 2021. Cet avis du HCSP alors conduit le gouvernement a préparé un arrêté visant la levée des restrictions. Les observations formulées ayant fait état dans leur grande majorité, de l'approbation des contributeurs concernant la levée des restrictions restrictions en vigueur l'arrêter a ici a été signé par les 4 ministères concernés et sa publication est désormais imminente. Je vous remercie. 43 secondes. Je souhaite simplement que la publication soit rapide elle aux fonctionnaires sont rapides pour poser des contraintes beaucoup moins rapide pour les lever. Merci la parole est à monsieur Marc que Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question concerne l'éligibilité. À la dotation politique de la ville. Concernant la la ville de Sedan 2ème commune des Ardennes après Charleville-Mézières et c'est un chef-lieu d'arrondissement. En effet depuis 2021 cette. Ville n'est plus éligible à la perception de la dotation politique de la ville du fait de l'absence de convention avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Sur cette politique. Toutefois, le centre ancien de la ville est reconnu comme quartiers prioritaires de la ville et ce en bénéficie d'une convention Agence nationale de rénovation urbaine dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. 2014 2024 pour la déclinaison du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. De plus, l'intégration du quartier le lac et son Transilien. Dans la liste des quartiers qui présentent des dysfonctionnements urbains les plus importants tels que est demandé permettrait à la ville de Sedan de figurer parmi les communes éligibles à la DPV compte tenu des enjeux démographiques socio-économique et financier. Je me permets de. Vous soumettre, de bien vouloir reconsidérer l'éligibilité de la ville de Sedan au dispositif de la DPV, telle que prévue à l'article 23 elle 23 34 tirs 40 du code général des collectivités territoriales notamment modifié par la loi de finances pour 2023, c'était l'accession à la DPV aurait. a fait un effet cumulatif avec le dispositif spécifique pact Ardennes qui vise à mettre en cohérence les politiques d'accompagnement social et urbaines pour renforcer l'attractivité du département des Ardennes. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Marc Laménie. La commune de Sedan. N'est effectivement plus éligibles à la dotation de politique de la ville, la DPV depuis 2021, a elle ne remplit plus plus l'un des 3 critères d'éligibilité prévu par la loi la convention ANRU dont elle disposait otite du 1er programme national de renouvellement urbain institué par la loi du premier août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et qui prévoit un effort national de transformation des quartiers les plus fragiles. En matière de logement, d'équipements publics et d'aménagement urbain a expiré. Vous le savez en 2019. Sedan a donc perdu sa DPV en 2021. La convention que vous évoquez qui porte sur le centre ancien de de Sedan relève d'un autre programme porté par l'ANRU le PNR quad qui a pour objectif de lutter contre l'habitat indigne dans les quartiers de centre-ancien et non dans les quartiers en politique de la ville. Elle ne permettent donc pas de bénéficier non plus de la DPV, la commune de Sedan et elle le sait peut néanmoins accéder à d'autres financements pour développer ses projets d'investissement au titre de la décide de la DETR ou du nouveau Fonds Vert mis en place par la Première ministre. Elle a également bénéficié des hausses de dotation de solidarité urbaine et rurale déçu et DSR prévus chaque année par les lois de finances depuis 2017 ça DGF a ainsi progressé de 158.415 euros entre 2017 et 2022 et représente désormais. Une capacité pour la ville de Sedan de 100 577 euros par habitant contre 164 euros en moyenne pour l'ensemble des communes. Cette hausse devrait se poursuivre en 2023 grâce à l'amendement par l'état des dotations de péréquation communal à hauteur de 200 millions d'euros pour la DSR et pour la DSR et 90 millions pour la DSU, je vous remercie. Merci monsieur Laménie vous n'avez que 6 secondes. Vous pouvez dire merci à monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Ministre, depuis on souhaite que je dirais ça va ça aille dans le bon sens pour la ville de Sedan, merci. Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à monsieur Jean Michel Arnaud. Merci madame présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi du 7 août 2015, la loi notre a rendu obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement des communes au comité de communes au comité d'agglomération au 1er janvier 2020, Un report jusqu'en 2026 a été produit est possible pour les comités de communes. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre, compte tenu. De la demande forte notamment dans les territoires ruraux et de montagne mais pas que dans un grand nombre de territoires de France, allez-vous enfin accepter l'idée. Que nous puissions avoir la liberté de choix d'exercice cette compétence dans le cadre communal et ou intercommunal à la main des communes. J'attends votre réponse avec beaucoup d'attention. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Sénateur Jean Michel Arnaud et. Je salue notre jeune public. Je n'ai pas encore vu je je rappelle que ce transfert a été décidé par la loi notre du 14 juillet 2015 pour 2020. Cette obligation a depuis été assouplies. Avec une date limite désormais fixé à 2026. La poursuite de ce transfert est une volonté forte du gouvernement. Cette disposition est essentiel. L'émiettement des services est un facteur d'inefficacité, comme l'a déjà souligné la Cour des comptes, plus les services couvre une population importante meilleure et la connaissance du réseau, son rendement et sa gestion. Le transfert de compétences au niveau intercommunal permet donc de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers et humains afin d'assurer une meilleure maîtrise des infrastructures de distribution d'eau potable et d'assainissement, et donc un service durable et plus performant pour les usagers. La sécurisation de cet approvisionnement tant en quantité qu'en qualité nécessite des interconnexions qui se raisonne à l'échelle des bassins de vie, voire du département. Par ailleurs, nous avons trouvé ces dernières années des solutions qui permettent d'apporter des solutions à beaucoup de problèmes locaux, les collectivités peuvent ainsi garder un prix de l'eau individualisé par secteur lors de l'entrée dans le PCI. Il est possible de garder des syndicats, on en a parlé pour assurer la compétence eau et et assainissement des solutions ont été élaborés et le Sénat. Il y a très largement contribué. Ainsi, le gouvernement ne soutiendra pas un texte visant à revenir en arrière sur les transferts de compétences eau et assainissement. À l'occasion des travaux de planification écologique. Le comité national de l'eau a exprimé la nécessité d'une stabilité de la législation à ce sujet les reports successifs ayant entraîné une posture d'attentisme des collectivités récalcitrantes préjudiciable à la bonne gestion de l'eau, je vous remercie. Merci monsieur Arnaud il vous, vous avez une minute 17. Oui, monsieur le Ministre j'entends évidemment les arguments régulièrement. Par votre administration sur l'inefficacité de la gestion. Des communes rurales vis-à-vis de leurs services d'eau. Je pense qu'elles apprécieront votre réponse de vous parler de collectivités récalcitrantes. Le terme est quand même particulièrement violent quand il s'agit de parler de liberté locale, matin, midi et soir, le gouvernement nous annonce la nécessité de faire confiance aux collectivités locales. Le couple préfets maires et valoriser et vous nous parlez de récalcitrants. Je trouve que le mot est est extrêmement déplacé. Nous aurons l'occasion de toute façon, de revenir sur ce sujet, puisqu'il y a ici une constance dans cette maison des propositions parlementaires de loi celle. De notre collègue sénateur de l'Ardèche Mathieu Darnaud celle de Jean-Yves Roux dans quelques jours et peut-être même celle d'un éminent sénateur centriste. Prochainement, donc je crois que il faut écouter la président de la commune de la délégation des collectivités locales. Françoise Gatel, il faut écouter. Les 2 tiers des collectivités intercommunales qui aujourd'hui écoute leurs communes membres et non pas décidé à ce jour de transférer la compétence. Oh, je crois qu'il faut effectivement que vous bougez de ligne. À défaut, ce sont les collectivités, les communes et les maires qui vous bougeront Monsieur le préfet, monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Salmon. Merci madame la présidente, monsieur le ministre ma question concerne le barème applicable aux articles de sports et de loisirs dans le cadre de l'arrêt du principe de responsabilité élargie du producteur, adoptée en 2020, la loi dit à Jacques à instaurer le principe de responsabilité élargie du producteur aux articles de sports et loisirs. Il n'est pas ici question de remettre en cause ce dispositif qui vise à renforcer l'effort de recyclage et à limiter à la source, la production de déchets. Cependant les critères retenus ne sont pas en adéquation avec les efforts réalisés par de nombreuses entreprises pour garantir la durabilité de leur produits. Un agrément a été confiée à la société écologique, qui a proposé un barème, basé sur les coûts réels de réemploi de collègues de dépollution et de traitement et incluant les fonds de réparation et de réemploi des articles de sports et loisirs cependant. Les barèmes retenu retiennent essentiellement le critère poids ce qui pénalise certains produits sans prise en compte de l'origine de leur cycle habilité ou de la valeur. À titre d'exemple un jeu de palets bretons composé d'une planche de bois et palais de fond est taxé à un euros 32 en 2023, 2 euros 22 en 2024 pour un produit fabriqué en France et vendu dans le commerce autour de 80 Un jeu de Cornol composé une planche de bois et de lui petits sacs en tissu rempli de grains et lui taxé à 2 euros 92 en 2023 et 4 euros 91 en 2024 pour un prix de vente lui aussi situé autour de 80 euros. À l'inverse, une table de billard composées de nombreux matériaux plus ou moins recyclable et taxé à 3 euros 18 en 2023 et 5 euros 34 en 2024 pour une valeur pouvant aussi là aussi les pour ce cas de 1000 euros à plusieurs milliers d'euros. Cette situation place plusieurs entreprises dans la difficulté. À titre d'exemple, une entreprise familiale bretonne utilisant des processus de fabrication, respectueux de l'environnement se voir redevable de 55.000 euros au titre de la crêpe. Pour 2022, sur un résultat de 150.000 euros en raison du poids de ces produits constitués de bois de fonte Matériaux pourtant reconnus pour leur durabilité, il me semble urgent de revoir ses barèmes pour les rendre plus cohérent et je souhaiterais donc connaître. Vos intentions sur ce sujet. Merci. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente. Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Daniel Salmon. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 à créer une nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur-REP pour les articles de sport et de loisirs. Chaque année ce sont 200.000 tonnes d'articles de sport et de loisirs neuf qui sont mis sur le marché. Sans filières REP ce sont autant de produits usagés qui seraient sans solution de réemploi ou de recyclage et qui finirait par être envoyés en décharge. Cette nouvelle filière REP a été lancée en 2022 et l'État a chargé un éco-, organisme d'organiser la collecte des produits usagés de financer les associations qui répare ses produits pour leur donner une seconde vie. Et de développer le recyclage des matériaux. Pour financer cette filière les fabricants et importateurs de produits neufs verse une contribution à cet éco-organisme pour couvrir les coûts de la collecte du transport et du recyclage des déchets. Ces coûts dépendent principalement du poids. Des déchets et de la valeur résiduelle des matériaux. La loi anti-gaspillage a également prévu des bonus et malus d'éco-conception en plus de cette éco-contribution. Il s'agit notamment de valoriser les critères de performance environnementale que vous évoquez comme la durabilité et la recycle habilité des produits. La feuille de route fixée à l'éco-, organisme prévoit d'étudier comment mesurer et valoriser ces 2 critères puis de proposer en conséquence des bonus malus d'IFSI fin 2024. Nous serons attentifs à ce que ces critères soient valorisés. Avec ses bonus et malus prévu par la loi anti-gaspillage pour favoriser des produits durables et recyclables. Je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Philippe Tabarot. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Un projet d'extension démesurée de la ferme aquacole située dans la baie de Golfe-Juan est en cours d'instruction. La préfecture des Alpes Alpes-Maritimes. Il est prévu de regrouper 3 concessions et par déjà existantes, en une structure dont les dimensions équivaudrait à 3 stades de football en surface et 15 sur le fond cette gigas structure de 24.000 m2 prévoit de passer sa production de 570 tonnes à 1200 tonnes par an. C'est un projet démultiplier qui questionne sur la qualité des eaux, la biodiversité les habitats naturels et potentiellement plusieurs espèces protégées dès la connaissance du projet les prud'homie des pêcheurs professionnels de Golfe-Juan, Antibes et Cannes ont lancé l'alerte très vite rejointe par les professionnels de la mer, la municipalité de Vallauris Golfe-Juan les plaisanciers les riverains pour s'opposer non pas l'aquaculture, mais à ce projet pharaonique. Nous étions encore vendredi dernier sur site, et nous sommes nombreux nous inquiéter de cette extension piscicole. Nous craignons des conséquences qui serait désastreuse en termes d'écologie qui contreviendraient aux impératifs de protection découlant du classement de la baie de Golfe-Juan. En zone Natura 2000 mais également en termes d'attractivité touristique et de sécurité de circulation maritime. Alors que l'enquête publique est en cours, l'État se prononcera-t-il concrètement contre cette autorisation. Alors que le maire de Vallauris ce sans spectateurs malgré lui, d'un projet d'implantation, pourtant rejeté par la population et sans même y avoir été associée en amont. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Philippe Tabarot. Tout d'abord je tiens à vous repréciser que l'enquête publique pour la procédure de concession sur le domaine public maritime est achevée depuis le 6 février, celle, celle portant sur l'étude d'un Pack et l'autorisation environnementale se terminera elle le 22 février. Les décisions à prendre, relève, vous le savez, de l'autorité du préfet de département. À l'issue de l'ensemble des procédures liées au projet et dans le cas où il serait donné droit à la demande de création de ce nouveau site les autorisations devront être assortie de prescriptions environnementales permettant bien sûr de respecter les écosystèmes marins. L'instruction par les services de l'État permet de s'assurer que le projet peut se développer en conformité avec les objectifs de conservation mais également en cohérence avec le schéma régional de développement de l'aquaculture marine et le document stratégique de façade Méditerranée dont le plan d'action a été adopté par les préfets coordonnateurs le 28 avril 2022. Le périmètre de 24.000 m2 que vous évoquez correspond au périmètre balisé désamarrage de surface des cages. Le volume de 1200 tonnes que vous évoquez aussi correspond au tonnage total de la production espérée par l'entreprise sur l'ensemble de son parc aquacole du littéral des Alpes Maritimes. Le projet est implanté dans un secteur identifié comme propice depuis 2015 dans le schéma régional de développement de la loi de l'aquaculture marine. Le projet prévoit en compensation, la fermeture de 3 sites existants représentant une surface totale de 6000 m2 et un potentiel total de production de 400 tonnes par an. L'État joue donc pleinement son rôle afin de garantir le respect de toutes les exigences environnementales et des échanges ont lieu régulièrement entre l'État, le préfet et ses services ainsi que les collectivités et les acteurs concernés. Je vous remercie. Merci mais Tabarot. Vous avez 25 secondes. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, votre réponse est inquiétante. Je le regrette. Au regard de la démesure prévisible des rejets de la pisciculture. Un projet qui détruirait des années d'efforts pour préserver la faune et la flore marine méditerranéenne et que vous allez semble-t-il cautionné. Merci la parole est à monsieur le président, Christian Cambon. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Un terrain de 10 hectares de friches industrielles sépare actuellement Paris et sa banlieue Est au niveau de la commune de Charenton, dont je salue le maire présent séance en 2016 un contrat d'intérêt national, a été signé entre cette ville de Charenton, l'État et le territoire Paris-Est Marne boit ainsi que Grand Paris Aménagement et la SNCF pour un travail collaboratif qui vise à créer un quartier qui va enfin gommé cette fracture urbaine. Un projet partenarial d'aménagement a été signé et au terme d'un appel d'offres à projets inventons la métropole du Grand Paris que vous connaissez bien Bouygues Immobilier a été désigné en 2018 lauréat de ce projet métropolitain. D'ores et déjà plus d'1.600.000 euros ont été dépensés. En études. Il s'agit de réaliser un programme très important 1600 logements, dont 30% de logements sociaux, des logements affectés à des des catégories particulières jeunes notamment étudiants et des bureaux, des commerces, des, des hôtels, des équipements publics avec, à la craie à la, à la clé la création de 15.000 emplois et bien évidemment, l'objectif est de redynamiser une partie de ce territoire en déclin et de réduire la coupure urbaine des entreprises ferroviaires entre Charenton nord et sud, tout en respectant les exigences de la SNCF. Nous en sommes aujourd'hui au dépôt du permis de construire, il faut donc que la SNCF formalise son accord car une partie d'un important du projet est assise sur les fonciers en sur sol des voies de chemin de fer. La SNCF a du reste été totalement associés l'instruction de ce projet. Or, en dépit d'un accord début 2022 en présence du préfet de région, excusez du peu. La SNCF vient de faire volte-face de manière assez Cavaliere et propose de décaler le permis de construire de 2 à 3 ans au motif qu'elle a des études complémentaires. Le amener. Alors Monsieur le Ministre, après 6 ans de négociations. Quelles mesures le gouvernement souhaite prendre pour ramener la SNCF a raison et ainsi offrir une belle opportunité de restructuration à un des derniers grands terrains de la métropole. Merci. Si la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Mais merci madame la la présidente mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président. Christian Cambon. Monsieur le maire que je salue. À mon tour le projet Charenton Bercy est une opération d'aménagement de grande ampleur dans le cadre d'inventons la métropole PREV. Permettant la création d'un nouveau quartier mixte comme vous l'avez rappelé, composé de 1600 logements, dont 30% de logements de logements sociaux vous imaginer à quel point le ministre de la ville et du logement. Il est aussi attaché. Ce projet permet aussi une nouvelle couture urbaine entre Charenton et la ville de Paris un désenclavement nécessaires et une requalification du secteur en écho au projet parisien Bercy Charenton. Le soutien de l'État à ce projet depuis plusieurs années, s'est manifestée en particulier par la prise d'initiative de Grand Paris Aménagement par la signature d'un contrat d'intérêt national en 2016 et par la qualification de grandes opérations d'urbanisme en 2021. Il se développe sur une dalle a réalisé en sur. Plon de foncier de la SNCF. Le dépôt de permis de construire de Bouygues requiert comme vous l'indiquez l'autorisation de la SNCF en qualité de propriétaire d'une partie des volumes foncier. La SNCF se préoccupe à juste titre des impacts de ce projet sur l'exploitation ferroviaire en particulier avec les fonctionnalités de la base de maintenance de l'axe Paris-Sud-Est. À terme et pendant la phase de travaux indépendamment des besoins d'exploitation. Le projet doit également composer avec la réalisation de voies de fret pour le futur hôtel logistique parisien qui crée de fortes contraintes. Ce projet, vous pouvez en être certain est suivie avec attention par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et par mon propre ministère délégué à la ville et au logement par le préfet de région Île-de-France en lien avec l'ensemble des parties prenantes concernées au cours des dernières semaines un important travail technique a été réalisé pour trouver un compromis satisfaisant chacun en associant bien évidemment étroitement la SNCF des discussions se poursuivent avec le ministre Christophe Béchu et et mes équipes et il réunira prochainement les principaux acteurs de ce dossier, je vous remercie. 3 secondes. Juste pour remercier le ministre de mettre toute sa volonté toute son action pour débloquer cette opération dans l'Est parisien bien besoin. Merci madame la. Et les trois secondes était en plus monsieur le président. Oui oui mais en plus. Non c'est pas ça si que vous aviez dépassé votre temps de 3 secondes. La parole est à madame Christine Bonfanti Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, en 2014, l'Union européenne avait adopté une directive de contrôle de véhicule motorisé cylindrée supérieure à 125 centimètres cube avec un objectif affiché de diviser par 2 en 10 ans le nombre de morts sur les routes. Le contrôle technique pour les deux-roues devrait ainsi selon une obligation européenne s'appliquer au plus tard au 1er janvier 2022 mais le gouvernement avait décidé, à juste titre de reporter cette obligation Anne 2023. Or, le 31 octobre 2022. Le Conseil d'État a annulé pour excès de pouvoir. Ce décret du 27 juillet. Il précise toutefois dans sa décision que la transposition effective de cette directive peut faire l'objet de mesures d'application différenciée. Ainsi le gouvernement bénéficie encore d'une marge de manoeuvre. Dans l'élaboration de ce contrôle. Rappelons qu'en France le pourcentage d'accidents des deux-roues qui sont liés à des défaillances techniques n'est que de 0 3 %. Tout le monde comprendra alors que le contrôle technique obligatoire n'est absolument pas une solution pertinente. Dans ce contexte européenne coercitif. Comment comptez-vous Monsieur le Ministre ne pas imposer le contrôle technique des deux-roues, tout en prenant en compte des remarques du Conseil d'État qui permettrait d'assouplir cette règle. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, madame. La sénatrice Christine Bonfanti Dossat. 2045 prévoit en effet qu'un contrôle technique périodique des véhicules à 2 roues motorisés de cylindrée supérieure à 125 cm3 soit mise en place à partir du 1er janvier 2022. Sauf si les États membres peuvent démontrer qu'ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les 5 dernières années.

Cependant à la suite de plusieurs procédures contentieuses initiée par des associations environnementales, le Conseil d'État a jugé que de telles mesures ne peuvent être regardées comme trop ponctuels et manifestement insuffisantes pour assurer efficacement la sécurité des usagers. Le gouvernement a donc pris acte de la décision du Conseil d'État. Toutefois, il faut souligner que cette décision ne conduit pas à une entrée en vigueur immédiate du contrôle technique, compte tenu de la nécessité de publier préalablement des textes d'application du décret du 9 août 2021, qui est celui, mettant en place le contrôle en vue de déterminer ses modalités de mise en oeuvre. Une consultation a donc été lancée en novembre par le ministre chargé des Transports, avec les associations de motards des associations environnementales et les représentants des professionnels du contrôle technique. Celle-ci a pour objectif d'identifier une solution acceptable pour tous dans le respect de la réglementation européenne le gouvernement veillera à tenir informer la représentation nationale des résultats de ces échanges. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre Madame Bonfanti Dossat vous avez 31 secondes. Merci Monsieur le Ministre. Mais je crois que d'autres solutions alternatives peuvent être encore. Et les motards sont prêts à travailler. Avez-vous pour les renforcer. Merci la parole est à monsieur Sébastien Pla. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Par l'arrêté du 31 décembre dernier qui instaure une taxe spéciale d'équipement pour contribuer au financement du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest vous infliger à 88 communes de l'agglomération de Carcassonne des communautés de communes de Castel. Castelnaudary l'Lauragais piège Lauragais ma Lepère une double peine, car les élus au droit du conseil départemental de ces agglo et des communautés de communes se sont déjà engagés à participer financièrement au financement de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ce chaînon manquant. Est ultra prioritaire pour notre écosystème économique et d'intérêt européenne majeure. Monsieur le ministre, je vous invite si vous le souhaitez, à prendre avec moi le, la LGV à Perpignan et vous verrez que nous irons plus vite pour rallier Madrid que pour venir ici au Sénat. C'est dire l'importance de ce projet. Monsieur le Ministre. Voilà qu'aujourd'hui le gouvernement nous impose de participer au bouclage financier du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest dont nous ignorons dans quelles conditions la liaison Toulouse-Narbonne elle verra le jour. Michael en quelque sorte vous nous proposer de payer pour voir. Je déplore que le ministère des Transports avant la promulgation du décret est ignoré mes nombreuses alertes ainsi que celles et ceux des élus locaux du risque induit par le choix du mode de calcul de la participation au financement. La facture risque d'être salée pour les communes situées à moins de 60 minutes d'une gare desservie par une future ligne à grande vitesse. Ce dispositif place l'ouest audois, dans l'obligation de financer les 2 projets de lignes à grande vitesse, c'est quelque chose c'est en quelque sorte la double peine pour eux. Alors si je souscris parfaitement au montage collective du financement des grands équipements structurants en faisant appel à la participation des collectivités locales concernées. Je ne peux accepter cette injustice qui frapper des collectivités certes volontaire mais aux moyens limités, pouvez-vous prendre l'engagement que des ajustements vont être proposées afin d'éviter aux habitants de ce territoire comme aux entreprises d'être doublement assujettis au financement des grandes infrastructures ferroviaires. Merci. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Sébastien Pla. Afin d'alléger la contribution budgétaire des collectivités territoriales dans le financement du grand projet ferroviaire Sud-Ouest. GPS ou une taxe spéciale d'équipement, vous l'avez rappelé a été institué dans la loi de finances pour 2022 dans les communes situées à moins de 60 minutes en voiture des gares desservies par le projet. Certaines communes de l'ouest audois, sont concernés par cette taxe à l'initiative des collectivités territoriales, des amendements à la loi de finances pour 2023 ont été adoptés par le Sénat et viennent compléter ce dispositif en instituant notamment une taxe additionnelle à la taxe de séjour affecté au financement du GPSO mais également dans la nouvelle ligne Montpellier Perpignan L N MP à partir de 2024, ce dispositif distingue un périmètre pour chacun des 2 projets ainsi les recettes perçues à ce titre dans le département de l'Aude bénéficie à la seule société de la LNM Certains contribuables de l'Est au doigt à moins de 60 minutes de Toulouse sont donc assujetties à la taxe spéciale d'équipement au bénéfice du GPSO. Les visiteurs et touristes de ces territoires seront quant à eux, concernés par la taxe additionnelle à la taxe de séjour au titre de la LNM. Néanmoins, les contribuables de l'ouest audois, ne sont pas davantage abs imposer que leur homologues concernés par ces taxes notamment l'Est de la Haute-Garonne et l'ouest audois, sont soumis à la même fiscalité si ce n'est que la surtaxe de séjour est perçue au profit de la LNM. Dans l'Aude et au profit du GPSO dans la Haute-Garonne. Je vous remercie. Merci Monsieur plats vous avez 14 secondes. Monsieur le Ministre, ne prend pas la même chose. Une taxe additionnelle à la taxe de séjour est payé par les touristes qui viennent sur le territoire alors que la taxe. D'équipements et est financé par les contribuables du territoire donc c'est pas la même chose Les touristes payeront certes partout sur l'ensemble du territoire départemental mais dans l'ouest audois, à cause de la taxe locale d'équipement. Ce sont une double imposition que les contribuables et les entreprises vont devoir payer. Merci la parole est à monsieur Daniel Laurent. Madame la présidente, monsieur le ministre ma question porte aussi sur la taxe spéciale d'équipement grand projet ferroviaire Sud-Ouest introduite dans la loi de finances par le gouvernement. Pour 2022, pour financer l'aménagement des lignes à grande vitesse Bordeaux Toulouse Dax. Ce n'est qu'à la publication de l'arrêté du 31 décembre 2022, établissant la liste des communes que nombre d'entre elles ont pris connaissance qu'elles étaient concernés. Dans mon département. Cette taxe s'appliquera dans 67 communes au motif qu'elles sont situées comme les 2342 autres à 60 minutes par véhicule d'une guerre desservie par la LGV. Si vous êtes à 61 minutes vous y échapper. Quelle logique d'équité. Quand vous connaissez les conditions de circulation pour atteindre la métropole bordelaise c'est quasi mission impossible pour nombre d'entre elles. Cette mesure a révolté élus mobilisés depuis plusieurs années sur la question des nuisances générées auprès des riverains par la LGV Sud Europe Atlantique sans parler de l'absence de travaux de maintenance toujours pas financé sur l'axe Nantes-Bordeaux qui génère un allongement des temps de parcours et une qualité de service moindre alors que la fracture territoriale en termes de mobilité est une réalité dans les territoires ruraux et périphériques des métropoles, vous comprendrez aisément les réactions proposée par ceux provoqués par cette mesure. Après la crise sanitaire. Un contexte international incertain, un taux d'inflation qui obère les finances des ménages, ce prélèvement supplémentaire pèsera sur les propriétaires et les entreprises. C'est inadmissible et inéquitable. En conséquence, Monsieur le Ministre, quelles réponses pouvez-vous apporter aux élus, aux administrés et aux entreprises qui vont devoir payer pendant 40 ans une taxe annuelle estimée pour le moment, entre 4 et 8 euros. Merci. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Daniel Laurent. À la demande des régions Nouvelle Aquitaine. Et Occitanie. Le gouvernement a créé par ordonnance en application de l'article IV de la loi d'orientation des mobilités. La société du grand projet du Sud-Ouest, établissement public local visant à faciliter le financement de ce projet par les collectivités via la mobilisation de ressources fiscales dédié. Comme vous l'indiquez afin d'alléger la contribution budgétaire des collectivités territoriales et à leur instigation, une taxe spéciale d'équipement a été instituée au profit de la société de projet dans la loi de finances pour 2022, à hauteur de 24 millions d'euros. Dans les communes situées à moins de 60 minutes en voiture des gares desservies par le projet. Ce dispositif a par ailleurs été conforté est complété par un amendement sénatorial dans la loi de finances 2023. L'arrêté du 31 décembre 2022 vient permettre la mise en oeuvre de ces dispositions législatives en précisant la liste des communes assujetties conformément à la méthodologie prévu par la loi de finances pour 2022 et et donc connu depuis plus d'un an. De ce fait, les contribuables de certaines communes de Charente-Maritime situé à moins de 60 minutes de la gare de Bordeaux sont assujettis à cette taxe. Il convient toutefois de souligner que le dispositif prend en compte le contexte actuel en limitant l'effort financier des contribuables. La société du GPSO a en particulier indiqué que le montant pour le propriétaire d'bien d'une valeur locative de 1000 euros serait de moins de trois. 3 cinq euros en 2023. Je vous remercie. Merci monsieur Laurent. Vous avez 18 secondes. Si madame la présidente. Tout simplement vous dire Monsieur le Ministre, cette injustice parce que je considère que nous sommes égaux sur un territoire. Nous devons profiter des mêmes équipements et c'est l'État, les collectivités auprès de qui nous payons des impôts qui doivent entreprendre ces investissements et et donc pas des gens ciblés sur un territoire à 60 minutes ça ne correspond pas du tout à la réalité. Merci d'en tenir compte. Merci la parole est à madame Nadia Sollogoub. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur la situation de la ligne trains d'équilibre du territoire TNT Paris-Clermont-Ferrand qui dessert la gare de Nevers dans la Nièvre les trains au départ de Nevers en direction de Paris n'ont pas pas d'itinéraire alternatif sauf être détourné vers 5S. Depuis 9h, ce qui occasionne une heure de trajet supplémentaires à minima pour éviter le secteur de Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne, qui constitue un véritable goulot d'étranglement sur ce tronçon très précisément les installations ferroviaires peuvent permettre en cas de besoin. La circulation d'un train en sens contraire mais sous réserve d'une procédure manuelle peu performante en matière de débit sur ce même tronçon les trains TNT subissent le trafic des trains de banlieue qui ne peuvent pas être dépassé sauf en gare. Ces constats appellent la nécessité de procéder à des aménagements des voies à Moret-sur-Loing, notamment pour améliorer l'insertion des trains qui desservent la Nièvre. Par ailleurs, suite à la Citura saturation du trafic en gare de Lyon depuis des années les trains qui desservent la Nièvre. Sont partent et arrivent maintenant gare de Paris-. Bercy mais face aux limites des infrastructures en place une amélioration du trafic serait souhaitable par la création d'un saut de mouton travaux réalisable sans interruption du trafic et qui permettrait de participer fortement à la limitation de ce phénomène de retards en cascade qui affecte l'ensemble des trains qui circulent sur cette ligne, je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, Nadia, Nadia pardon ce logo. Je vous confirme que la modernisation de la ligne Paris-Clermont-Ferrand fait partie des réalisations prioritaires de l'État en matière de modernisation des lignes existantes. Ligne sur laquelle le ministre chargé des Transports a lancé un groupe de travail le 15 septembre dernier, Poursuivre l'amélioration de la qualité de service, en plus du comité de suivi annuel. L'infrastructure de la ligne fait depuis plusieurs années, l'objet d'investissements conséquents dans le cadre du schéma directeur de la ligne approuvé par l'État en 1er lieu un programme de régénération de l'axe pour lequel SNCF réseau investira 760 millions d'euros jusqu'en 2025 et lancé la trajectoire prévisionnelle est aujourd'hui tenu malgré la crise sanitaire. D'autre part, un programme de modernisation à la hauteur de 130 millions d'euros cofinancés par l'État et la région. Auvergne-Rhône-Alpes est en préparation. Enfin le schéma directeur prévoit également l'arrivée de nouveaux matériels roulants qui représente un investissement de 250 millions d'euros pour les rames qui circuleront sur cette ligne. Ces investissements permettront une amélioration de la robustesse d'exploitation sur l'ensemble de la ligne perd on perd Paris Clermont, y compris pour la desserte de la Nièvre. Comme vous le savez l'actualisation de la programmation pluriannuelle des investissements dans le domaine des transports est actuellement en cours de préparation. Le rapport du conseil d'orientation des infrastructures préparé à cet effet sera prochainement remis à madame, la Première ministre. Le financement et les conditions de poursuit des études jusqu'à l'enquête publique pourront être discutés avec les co-financeurs du projet et en particulier la région Île-de-France, je vous remercie. Merci, même sur le groupe, vous avez 37 secondes. Oui, je vous remercie Monsieur le Ministre, je sais qu'il y a des travaux qui sont prévus et vous me parlez de changement des rames, mais moi je vous parle de saturation de la ligne d'autant plus qu'il y a les trains également TER qui desserve cours de Paris il y a dans la Nièvre, des gens qui font tous les jours depuis 2 au comme la liaison avec Paris, ils sont saturés, saturés, excédés, ça devient totalement insupportable, parce que les dysfonctionnements sont maintenant quotidien il faut il faut vraiment prendre ce situation en compte parce que ils n'ont pas d'autre solution maintenant que de prendre la voiture finalement les trains d'équilibre des territoires sont un train déséquilibré qui déséquilibre notre territoire. Je vous remercie. Merci la parole est à madame Annick Jacquemet. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la responsabilité des maires en cas d'agression, de personnes d'accident ou d'atteintes aux biens, à la suite d'une interruption volontaire de l'éclairage public. Je viens de terminer un rapport pour l'OPEP sur la pollution lumineuse, dont les conclusions invite notamment les mères à produire un effort de sobriété lumineuse et énergétique raisonner en matière d'éclairage public plusieurs raisons légitimes peuvent être invoquées pour justifier une telle recommandation. D'abord les défis liés à la transition écologique, puisque dans notre pays, le seul éclairage public et mais 670.000 tonnes de CO2 par an, ensuite les réelles préoccupations sur la santé publique, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes ou sur la biodiversité engendrée notamment par l'utilisation des LED. Enfin, l'éclairage public représente en moyenne 41% de la consommation électrique des communes dans le contexte de crise énergétique et compte tenu de la flambée des coûts, l'électricité, la modulation de l'éclairage public constitue pour elle une source d'économies budgétaires importantes. De nombreux élus d'ores et déjà sensibilisé à ces enjeux ont commencé à agir. Près de 12.000 communes ont fait le choix de réduire voire supprimer l'éclairage public la nuit. Le problème c'est qu'aujourd'hui ce sont potentiellement 12.000 maires qui prennent des risques, puisqu'en l'état actuel du droit. Ces derniers ne sont pas suffisamment protégés. En effet, même si le juge administratif admet que chaque maire puisse fixer volontairement des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit. Sa responsabilité est susceptible d'être engagée en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire claire. Ainsi, au regard des enjeux évoqués de l'inquiétude des maires concernés. Quelles sont les intentions du gouvernement pour définir ce cadre législatif et réglementaire autour de cette question et sous quel délai, je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente. Merci, peut-être pour la dernière fois aujourd'hui. Mesdames, ces messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, Annick. Jacquemet. Merci pour votre question. Et je rajouterai un sujet le professeur de physique chimie, que je suis grand âne amateur d'astronomie confirme l'intérêt de lutter contre les pollutions lumineuses le le juge administratif examine en en cas, au cas par cas, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutif d'une carence du gestionnaires de voirie et ou du maire susceptible d'engager la responsabilité administrative des collectivités Au delà de l'intervention du juge administratif la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police peut aussi conduire à la constitution d'infraction susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Même si cela paraît limité. En effet, si l'absence d'éclairage public était considéré comme directement à l'origine du dommage la responsabilité du maire ne serait susceptible d'être engagée qu'à la condition qu'il n'est pas accompli les diligences dite normale au sens de l'article L 21 23 34 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le dommage est indirecte, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l'article 121 3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, que le maire ne pouvait ignorer parce conséquent les infractions d'homicide ou de blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que maire c'était délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique. Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré. Le gouvernement ne compte pas faire évoluer le cadre juridique des responsabilités administratives et pénales des maires et des collectivités territoriales en matière d'éclairage public, je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Ministre quand la gestion de du temps. Merci beaucoup. La parole est à madame Chantal de scène. Merci madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur l'augmentation importante du nombre d'annulations de rendez-vous médicaux à la dernière minute au détriment du temps médical destiné à la population et ce dans un climat de tension et de difficulté d'accès aux soins chaque année près de 27 millions de rendez vous ne sont pas honorés. C'est insupportable pour les médecins et les patients qui attendent un rendez-vous l'article R 41 27 tiré 53 du code de la santé publique, dispose que les honoraires ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectuées. Pour cette raison, il est interdit de facturer des honoraires de consultation. Si le patient ne se présente pas au rendez-vous. Pourtant dans des conditions strictes. On pourrait imaginer que le service de réservation et non celui de la consultation puisse faire l'objet d'une facturation afin de dissuader ces incivilités qui ne sont pas sans conséquences, une régulation financière. Pourrait être en place avec l'aide des plateformes de réservation. Une précision dans le code de la santé publique pourrait ouvrir la possibilité pour les professionnels de santé d'être dédommagés pour un temps médical qui leur a été soustrait. Madame la Ministre sur la base de cette proposition, je souhaiterais connaître les intentions du gouvernement sur ce problème. Merci la parole est à Mannheim Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Bonjour madame la ministre. Bonjour madame, merci madame la présidente, madame la sénatrice. Vous appelez mon attention sur l'augmentation importante du nombre d'annulations de rendez-vous médicaux à la dernière minute, voire sans prévenir au détriment du temps médical dans un climat de tension sur l'offre médicale et de difficultés d'accès aux soins alors de très nombreux soit sur le terrain, j'ai pu le remarquer, je partage votre préoccupation par rapport à ces créneaux bloqué en vain qui conduisent à gâcher un temps médical précieux alors que certains de nos concitoyens peinent à obtenir un rendez-vous lorsqu'ils en ont réellement besoin. À l'occasion de ses voeux aux acteurs de la santé, le président de la République a pris position en ce sens et a annoncé qu'un travail serait engagée avec l'assurance maladie pour supprimer cette perte sèche de temps médical et responsabiliser les patients lorsqu'un rendez vous où plusieurs ne sont pas honorés ou lorsqu'il y a des recours abusif à des soins non programmés. C'est dans cette logique de responsabilité collective, de droits et devoirs âgé que le ministère de la Santé Oeuvres de manière prioritaire à sensibiliser la population à cet enjeu qui nous concerne tous aussi avant d'envisager une pénalisation financière de ses patients. Il nous faut davantage réussir à objectiver la prévision de ce volume de rendez-vous non honorés. On parle de 28 millions. Mais rien n'est moins sûr, mais on sait mais on sait que c'est en fait, nous manquons en effet malheureusement à l'heure actuelle de données précises et partagé entre tous les acteurs. Une fois cet état des lieux établi, nous pourrons envisager différents nouveaux leviers pour réduire ce phénomène en lien avec toutes les parties prenantes. Mais je le dis à nos concitoyens le temps médical et précieux. Vous prenez un rendez-vous, respectez le. Merci. Même de scène. Vous avez 36 secondes. de pénurie de médecins d'avoir certains de nos concitoyens. Qui omettent d'annuler leurs rendez-vous. C'est inacceptable. Donc je compte sur le gouvernement pour mettre en place un dispositif pour responsabiliser éduquer les éventuels patients. Merci la parole est à madame Patricia de masse. Merci madame la présidente, madame la Ministre. Le maire de la commune de Puget-Théniers. Dans mon département des Alpes-Maritimes. Ah via le conseil départemental identifié une médecin de nationalité marocaine depuis déjà quelques mois pour lutter contre la désertification médicale qui frappe son territoire. Cette jeune médecin qui a obtenu son diplôme en Europe, en Espagne il y a quelques années à effectuer un stage en France émettrice donc parfaitement notre langue. Elle a de plus exprimé le souhait de s'installer dans ce territoire de la ruralité. Or le temps passe et le parcours administratif pour valider sa venue devient long et pourrait même finir par en être compromis naturellement la vérification des compétences est un absolu préalables, mais l'information sur les documents à produire et la procédure à suivre ne semble pas suffisamment connu par ailleurs les délais de vérification des documents semble anormalement long il en partie aussi de l'obtention de titre de séjour en préfecture encore que la possibilité de demander et d'obtenir rapidement des passeports talents soit désormais ouverte en théorie. Il en va surtout de la certification pour le CNG dans les délais d'instruction sont anormalement longs sans qu'on puisse comprendre ce qui justifié. Alors que les mesures activé par le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux tarde tu à produire des effets. Il est regrettable que ces lenteurs et obstacles de nature administrative pénalise l'installation rapide de médecins jusqu'à parfois l'en dissuader, je souhaiterais savoir Madame la Ministre si le gouvernement a bien pris toute la mesure de ses lenteurs. Si une communication pour mieux faire connaître les procédures ne pourrait pas être envisagée pour faciliter l'action des maires. S'il ne simplification surtout des procédures comme un raccourcissement des délais de traitement des candidatures par le CNG ne pourrait pas être prévue dans l'intérêt des collectivités. En manque cruel de médecins généralistes, particulièrement en zone rurale. Je vous remercie. Merci la parole est à Madame Agnès Firmin Bodo Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, l'autorisation d'exercice pour les praticiens à diplôme étranger, Union européenne et hors Union européenne est un enjeu individuel pour les intéressés mais aussi une mesure permettant de garantir le maintien d'une offre de soins dans de nombreux territoires comme vous venez de le signaler. La seule voie d'accès à l'autorisation d'exercice pour les pas du et la réussite aux épreuves anonymes de vérification des connaissances, les EVC organisée actuel annuellement par le CNG qui permettent de s'assurer des acquis fondamentaux et des connaissances pratiques, les lauréats doivent ensuite réaliser un parcours de consolidation des compétences de 2 années d'exercice en établissement pour obtenir leur l'autorisation de plein exercice salariées ou libérale pour obtenir de plus amples informations sur cette procédure les pas du et. Les élus peuvent se rapprocher des ARS, elles seront leur préciser les documents à réunir et pourront s'assurer que les médecins remplissent les conditions pour se présenter aux épreuves. Par ailleurs, dans le cadre du prochain PJ l'immigration il est envisagé de créer une carte de séjour pluriannuelle pour les professions médicales et de la pharmacie, connu sous le nom de passeports talents au début des travaux du gouvernement. Cela permettrait aux pas du qui ne auront pas encore la condition de l'obtention des. Et qui s'engagent à les passer mais qui satisfont aux critères nécessaires à l'obtention d'une attestation d'exercice provisoire de venir exercer en France sans attendre pour une durée limitée. Ce serait une mesure concrète pour les praticiens qui se trouve empêchée pour cette seule exigence de venir exercer en France ce sera également un levier d'attractivité pour tous les pas du en leur faisant bénéficier du dispositif avantageux des CSP talents dans l'objectif du fluidifier les parcours d'accès à l'exercice et de répondre à nos besoins de court terme en matière de professionnels de santé. Merci la parole est à monsieur Georges Patient. Ça va présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question est destinée au ministre de la Santé. À qui j'ai déjà adressé un courrier sur ce sujet. Courrier demeurées sans réponse à ce jour. Aussi Madame la Ministre je reviens une fois de plus alerter et vous sensibiliser sur l'état d'avancement du projet de CHU de Guyane. En effet l'objectif initial d'ouverture fixée au 1er janvier 2025 par vos collègues et prédécesseur semble compromis. Une situation forte inquiétante pour la population guyanaise, qui attendent depuis trop longtemps l'égal accès à la santé. La population guyanaise en a fait légitimement une priorité acté dans les accords de Guyane de 2017. Le gouvernement a pris la décision de création en mars 2021 mais depuis, force est de constater que le dossier n'avance guère. Certes on peut noter quelques avancées qui préfigure la création du CHU. Mais il existe surtout des dissensions, des blocages qui viennent freiner le Bonnafont suspendu projet voire interpelle sur la réelle volonté de tous les acteurs de créer ce CHU. Premièrement ce CHU a été conçu sur le pré de qui, d'une fusion administrative entre les trois centres hospitaliers de Guyane. Celle-ci est actuellement inopérante, faute de consensus. Qu'en est-il. D'autre part les formations pour le personnel nécessaire sont-elles mises en place sont-elles assurées. Devons-nous continuer à dépendre indéfiniment de la réserve nationale. Plus inquiétante encore, est la question du financement des nombreux chantiers il m'oublier notamment sur Cayenne et sur Kourou du matériel nécessaire pour la mise en place de ce CHU. D'après certaines estimations le besoin s'élèverait à 800 millions d'euros. Or à ce jour, rien n'a été arrêté concernant cette opération. Eu égard à la configuration du territoire au dynamisme démographique a l'effort massif de rattrapage a réalisé ce montant doit être allouée à la Guyane. À l'instar de ce qui a pu être fait pour d'autres territoires. Madame la ministre, le gouvernement entend-il en faire bénéficier la Guyane et quand ce montant sera-t-il matérialiser je vous remercie. Merci la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, le ministre François Braun regrette de ne pouvoir être présent ce matin il m'a prié de vous fournir les éléments suivants, en réponse à votre question. Comme vous le soulignez ce projet ambitieux. D'autres employes de l'offre de soins que de la formation et de la recherche reposant sur 4 piliers que sont les trois hôpitaux de Guyane et le réseau des CDPS. La première étape de ce projet consiste en la création de 3 hôpitaux de proximité. Et Marie pas pas sous la grand-senti et Saint-Georges de l'Oyapock. Cette première étape a grandement mobiliser les équipes qui malgré l'épidémie de code 1019 ont pu présenter en 2022, les 3 projets aboutis, lesquels ont ensuite fait l'objet de concertations nourries. Les autorisations de médecine ont été délivrés. Ces nouveaux hôpitaux pour lesquels des Travaux et recrutements sont en cours pourront ouvrir cette année c'est une avancée réelle pour les populations de ces territoires, elles pourront être hospitalisé pour de courts séjours de médecine au plus près de chez elle et bénéficieront d'une offre de radiologie et de biologie de proximité. La 2ème étape la plus structurante pour l'avenir est en cours, c'est celle conduisant à construire à conduire l'univers sa théorisation des hôpitaux du territoire et à conduire l'intégration du projet médical de formation et de recherche des établissements c'est ce projet qui sera le ciment des différents sites, qui réunira les équipes et les fera coopérer au mieux dans la construction de ce projet. Il est également nécessaire de séquencer les étapes. Le sujet du chantier administratif interviendra dans un second temps, une fois le projet finalisé et au service de celui-ci, il en va de même pour les projets d'investissements complémentaires à ceux déjà en cours qui ne sont pas un préalable mais des moyens de concrétiser le projet une fois celui-ci aboutit. Les équipes sont pleinement à l'oeuvre et les premières orientations médicales et de recherche semble partagée par tous, aussi je suis avec le ministre-confiantes dans leur capacité collective et grâce à l'engagement personnel du président, Gabriel Serville à aboutir à un projet de territoire permettant d'initier la dynamique d'université réalisation à horizon 2025. Merci la parole est à monsieur Alain Milon. Oui merci madame la présidente, madame la ministre je souhaite attirer votre attention sur l'inégalité de traitement dont sont victimes les établissements publics de santé et les établissements et services médico-sociaux publics en matière d'abattement de cotisations sociales pérennes. En effet, les pouvoirs publics ont décidé depuis 2019 d'accorder un abattement de cotisations sociales pérennes à l'ensemble des opérateurs privés. Cet abattement de cotisations représentent une réduction du coût de salariale d'environ 8% particulièrement stratégique dans le secteur de la santé et de l'autonomie ou la masse salariale représente jusqu'à 90% d'écoute pour autant le gouvernement a décidé d'en exclure les établissements publics de santé et les établissements et services médico-sociaux publics. Or, si dans le Champ sanitaire les établissements privés ont vu leurs tarifs réduits en compensation de la baisse de cotisations, rien de tel ne s'est produit dans le dans le secteur médico-social, au moment où les errements de certains groupes privés qui bénéficient de ces amendements de cotisations sociales ont été mises à jour il paraît impensable de continuer à taxer plus lourdement les établissements publics dont les Budgets sont eux intégralement contrôlé, vous le savez par les ARS et les conseils départementaux afin de mettre fin à cette inégalité de traitement et permettre aux ce SMS public de se moderniser, de recruter le personnel indispensable à la qualité d'accompagnement des usagers Madame la Ministre quelles dispositions du gouvernement entend-il, mettre en oeuvre et dans quel délai. Merci la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur. Cette réduction de 6 points du taux de cotisation d'assurance maladie est applicable depuis le 1er janvier 2019 aux entreprises du secteur privé. Elle s'est substituer Or les établissements publics ne bénéficiaient pas du CICE puisqu'ils ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la création de cette réduction n'a donc eu aucun effet sur l'équilibre de l'imposition sociale et fiscale entre les établissements publics et les établissements privés, de manière générale, le secteur public ne bénéficient pas des mêmes dispositifs d'exonérations que le privé puisqu'il n'est pas soumis au même régime de prélèvement par nature ces établissements sont pour la plus grande part financé par des ressources publiques. Il n'est pas possible de leur appliquer des raisonnements propre au secteur concurrentiel. Élargir le bénéfice du bandeau maladie de 6 aux ce SMS public reviendrait indirectement à augmenter le financement de ces structures par l'assurance maladie en diminuant des cotisations qui reviennent directement à cette branche le canal des exonérations des cotisations sociales n'est pas le plus approprié. Par ailleurs, je tiens à le rappeler. Le gouvernement est pleinement engagée dans le soutien de SMS avec des efforts conséquents réalisés en ce sens le Ségur de la santé a permis un financement exceptionnel d'un total de 2,1 milliards en 2021, 25 pour le soutien à l'investissement dans le secteur médico-social et a été prévu une revalorisation des rémunérations des personnels des établissements publics de santé et des pas de 183 euros Net a minima majorée pour les soignants. Cette revalorisation a été étendue aux autres SMS par la conférence des métiers du 18 février 2022, les Jeux SMS ont perçu plus de 3 milliards. une prime grand âge spécifique au secteur public a été créé en 2020 pour 161 millions d'euros. Je vous remercie. Merci Monsieur Mignon, vous avez 38 secondes.

qui a été cumulé durant les années précédentes, il n'est donc pas ici. Il n'entraîne pas obligatoirement de de conséquences pour le reste des établissements nous savons quand même que la tarification publique progressent beaucoup moins vite que l'État Que la tarification privée pardon et que le public comme le privé subit d'inflation, on constate donc une fragilisation masse majeur de l'offre publique médico-social et je vais peut être terminée par une phrase qui vous plaira peut-être pas. Il est grand temps Madame la Ministre de réagir pour favoriser la renaissance du public. Merci. La parole est à même la présidente Catherine Deroche. du nombre de cas d'infections invasives à méningocoques depuis la levée des gestes barrières. En 2021, avec une nette accélération de l'augmentation sur la fin d'année 2022, notamment chez des enfants jeunes, des adolescents et des adultes jeunes derrière ces chiffres, il y a des vies humaines. De nombreux cas tragiques ont été partagées par la presse et plusieurs ARS alerte sur des situations épidémiques, un enfant de 3 ans ainsi scolarisés dans une école d'Angers est décédé en octobre dernier d'une méningite de. Sérogroupe Y.. Cette situation épidémiologique doit conduire la HAS à revoir sa position concernant la recommandation vaccinale datant de mars 2021, quand l'épidémiologie des maladies infectieuses était ralentie du fait des mesures barrières. La solution existe. La simple substitution du vaccin. C'est par un vaccin ACW. Y permettrait de conserver un nombre de rendez-vous et d'injection constant d'un petite enfance mais à Valence accrue sans travail supplémentaire pour les professionnels de santé, vaccinés. il existe 3 vaccins ACW. Mais ils ne sont à ce jour ni recommandé ni remboursé pour l'ensemble des enfants. Il est donc nécessaire d'assurer la prise en charge par la solidarité nationale de ces vaccins dans un but de réduction des inégalités sociales de santé et je voudrais savoir Madame la Ministre on en est

Merci madame la présidente, madame la sénatrice. La situation épidémiologique des infections invasives à méningocoques fait l'objet d'une surveillance en temps réel et d'une vigilance élevée de la part du ministère de la santé de santé publique France 2 Centre national de référence, ainsi que de la HAS en charge des recommandations vaccinales nationale s'agissant des méningocoque du sérogroupe B, la vaccination de l'ensemble des nourrissons fait l'objet d'une nouvelle recommandation dans le calendrier vaccinal. 2022. Elle est ainsi depuis le mois d'avril 2022, prise en charge par l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres vaccins, s'agissant de la stratégie de vaccination contre les méningocoques A C W et Y la HAS avait rendu en a mis un avis en mars 2021 à cette époque en l'absence d'augmentation des infections. La vaccination de l'ensemble des nourrissons par le vaccins tétravalents couvrant les souches A C W Y n'avait pas été recommandé la HAS a toutefois indiqué qu'au regard de l'importante variabilité de l'épidémiologie des infections invasives à méningocoques une vigilance particulière était nécessaire pour évaluer la pertinence d'un futur élargissement de la vaccination méningocoque après plus des années de faible incidence notamment liées aux mesures sanitaires mises en place durant la pandémie de Covid-19, le nombre de cas d'infections connaît une nouvelle hausse depuis octobre 2022. Les cas sont en grande majorité liés au sérogroupe B 53% Y. 23% et W 19% en réponse à cette récente augmentation la HAS a repris ses travaux de révision de la stratégie 2021 de vaccination contre les infections invasives un méningocoque de manière globale. La recommandation actualisées seront mises en oeuvre dès leur publication par la chasse. Merci madame la présidente de Roche, vous avez 27 secondes. Je pense en effet que c'est un sujet important, j'étais jeudi à un colloque organisé par l'association Audrey qu'une association de mon département. Devenue association devenue méningite France Santé publique France a été très clair sur les cartes et notamment sur la France qui était un peu isolée avec ce vaccin. C'est alors que les autres pays européens. Étaient sur des des vaccins. Valant et et dans les mouvements, notamment des jeunes, des étudiants dans le cadre du programme Erasmus. On voit bien les risques que l'on fait peser, donc j'espère qu'en effet on pourrait arriver rapidement une solution. Merci la parole est à monsieur Éric Bocquet. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre la presse régionale des Hauts de France s'est récemment fait l'écho, les difficultés que rencontrent de nombreuses familles dont un enfant est atteint de troubles du spectre de l'autisme. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme 2018 2022 dans la région des Hauts-de-France diverses mesures ont été mises en oeuvre. À titre d'exemple, 999 enfants ont été intégrés au dispositif de plateformes de coordination et d'orientation et 1184 autres ont bénéficié d'une prise en charge. Ce dispositif constitue un Net progrès en matière de repérage et de diagnostic pour les enfants porteurs du trouble du spectre de l'autisme. Mais lorsque ces enfants grandissent et deviennent adultes. On constate qu'il y a un manque criant de structures prêtes à les accueillir. Pour pallier ce déficit de places depuis 1989 l'amendement dit amendement Creton, permet aux jeunes de 18 à 20 ans de rester en institut médico-éducatif faute de solution alternative. Or il apparaît que ces structures ne sont plus adaptés à leurs besoins et d'autres enfants plus jeunes attendent d'être pris en charge à leur tour de plus ils ne peuvent plus rester, on y est. Mais au-delà de 20 ans. Leurs familles se trouvent alors sans solution. Trop souvent, l'un des deux parents lorsque cela est possible doit cesser de travailler pour s'occuper à plein temps de son enfant, certes il est adulte mais il existe toujours une attention de chaque instant. Dans le département du Nord, les places en structure d'accueil pour les autistes adultes sont si peu nombreuses que les délais d'attente peuvent atteindre parfois plusieurs années. La situation qui était déjà tendu s'est encore aggravée après que l'Agence Régionale de Santé a pris la décision de ne plus financer les placements dans des établissements situés en Belgique où de nombreuses familles nordiste avait. Héberger leurs enfants auparavant laissant ainsi des familles démunies. Or il existe une solution des associations spécialisées sont prêtes à s'investir dans l'accueil. Une quarantaine de jeunes adultes pour peu qu'elle soit sollicités par un appel à projets de l'ARS des Hauts de France quel et madame le la vision et les solutions préconisées par le gouvernement sur ce sujet. Merci la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, la ministre Geneviève Darrieussecq regret de ne pouvoir être présente et m'a prié de vous fournir les éléments de réponse suivants à votre interrogation. L'autisme et les troubles du neuro-développement font partie des préoccupations majeures de nos politiques publiques. Les 490 millions d'euros qui ont été consacrés à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement en attestent. Pour la région des Hauts de France nous savons les besoins importants quelques données pour rappeler l'engagement de l'État ces dernières années. Création de 8 plateformes de coordination et d'orientation de 20 unités d'enseignement maternel autisme de 4 dispositifs d'autorégulation de 136 places pour personnes autistes et bientôt, création de 3 nouvelles unités de vie pour adultes autistes en situation complexe monsieur sénateur vous indiquer que l'ARS Hauts-de-France le finance plus l'accueil dans des établissements belges, permettez-moi de vous contredire sur ce point. Au 1er janvier 2022, 1508 adultes et 693 enfants du Nord voient leur accompagnement en Belgique financé par l'État français. Je le dis clairement, la France était en retard sur l'accompagnement des personnes autistes. Notre action ces dernières années permet de le rattraper. Les solutions d'accueil et d'accompagnement se sont multipliées pour autant toutes les personnes concernées ne trouve pas une solution satisfaisante, nous les entendons le cap est clair et l'engagement du gouvernement également être exemplaire. L'ouverture de la future Maison de l'autisme, voulue par le président de la République l'illustre parfaitement cette maison sera ressources pour les familles, encore trop souvent désemparés et permettra aux associations de se retrouver, d'avoir accès aux meilleures pratiques d'avoir accès à la connaissance de tous les aides et de tous les dispositifs. Elle permettra aussi de mieux faire comprendre ce qu'est l'autisme au plus grand nombre car il s'agit là aussi d'un enjeu essentiel. OK je sais ma collègue Geneviève Darrieussecq particulièrement attaché. Merci, madame la Ministre, la parole est à monsieur Max Brisson. Merci madame la présidente, madame la ministre, la production de laine de brebis des 3 races laitières présente autant d'épées l'Atlantique s'élève chaque année Hamilton si de petites entreprises en valorise une infime partie aucune solution n'existe pour la plus grande partie de la production. Pourtant, bien qu'elle ne soit pas adapté à certaines valorisations notamment textiles cette laine à de nombreux atouts reconnus. C'est pourquoi la chambre d'agriculture des pénates antique et la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ont initié un programme de recherche sur le traitement de la haine, achevée en 2022. 2 prototypes concluants ont été développés le compostage, qui permet aux éleveurs de valoriser la laine directement dans le, dans leur exploitation et de produire un compost plus riches pour leur prairie ou culture. La production de granulés fertilisant qui permet aux coopératives entreprises locales de commercialiser un Angry durable et locale à base de laine ces 2 prototypes s'ils étaient généralisée des débouchés intéressants pour la laine de brebis profitant à chacun des acteurs du secteur cependant leur mis sur pied bute sur des règlements européens. Résultat, bien que le processus de compostage permettent de lever des risques microbiologiques. Les conditions de sa réalisation sont rendus quasiment impossibles par la réglementation. Quant à la solution des granulés fertilisant, les éleveurs de mon département, constate que dans d'autres pays européens. Des entreprises et les commercialisent enfreignant ainsi la même législation européenne. Il en ressort alors une distorsion de concurrence inacceptable aussi Madame la Ministre ma question est simple, le gouvernement est-il prêt à soutenir la mise en oeuvre de ces prototypes innovants en engageant des négociations afin d'obtenir une évolution de la législation européenne. Merci la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, vous interrogez sur l'absence de débouchés pour la laine de brebis. Le ministère de l'Agriculture accompagne d'ores et déjà la filière ovine dans la structuration d'une filière laine à travers le plan d'action national bioéconomie, le plan de relance via le projet tricolore et la mise en place par FranceAgriMer d'un observatoire du marché des cuirs l'impôt et plume ainsi que d'un groupe de travail chargé d'identifier des pistes de valorisation pour ses productions. Concernant le volet sanitaire la laine a le statut de sous-produit animal de catégorie 3 au titre de la réglementation européenne pour cette catégorie des sous-produits animaux les possibilités de valorisation sont multiples et ouvertes à l'innovation, par exemple le textile. Les matériaux isolants, l'industrie pharmaceutique et cosmétique l'alimentation animale, les engrais néanmoins la réglementation européenne impose des règles pour son usage direct dans le sol en tant que fertilisant, compte tenu des risques sanitaires de diffusion de maladies animales pour les animaux d'élevage. La faune sauvage, voire pour l'homme. L'expérimentation Interreg potée fac Lana Allende présente un intérêt qu'il conviendra d'analyser avec attention la valorisation de la laine par le compostage sur place en élevage-elle autorisée mais nécessite l'obtention par l'établissement d'un agrément sanitaire couvrant la conformité des locaux des équipements et du fonctionnement ainsi que la sécurité et la maîtrise du procédé. Afin de faciliter les démarches des exploitants. La direction générale de l'alimentation à travailler avec la filière sur un dossier de demande d'agrément type pour les exploitants et à une flexibilité sur la fréquence des analyses d'auto-contrôle en complément, une mission du Conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux est en cours pour élaborer une feuille de route pour améliorer la valorisation et les débouchés de ces produits. Le rapport est attendu pour avril 2023. Si ma ma ministre monsieur Brisson. Vous avez 29 secondes. Merci madame la présidente, je vous remercie, madame la Ministre, pour ces précisions. Je crois que les professionnels et les deux chambres, salle d'agriculture et celle de commerce de commerce et d'industrie Pau Béarn attends deux rapidement ses analyses attends de cet agrément, cela pourrait constituer des débouchés réels qui apporterait des réponses aux éleveurs, aux entreprises, aux coopératives et aussi d'ailleurs aux deux chambres, qui ont beaucoup plus investi avec des soutiens comme vous l'avez dit du époque Taifa dans ces 2 prototypes qui mérite certainement une une analyse fine, être le plus vite possible référencés et agréés. Je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Jean-Yves Roux. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Les pommes des Alpes. D'autres provinces grâce à un ensoleillement exceptionnel et des variations de température qui favorise une bonne teneur en sucre et une acidité remarquables constitue une fierté pour notre département. Depuis 2018, les 250 exploitations agricoles qui produisent pour une grande part des Golden ainsi que des pommes Gala ont effectué un travail de diversification importante pour s'adapter à des embargos russes, chinois et algérien ainsi qu'à des iPod des épisodes de grêle et de gel répéter. Aujourd'hui ces arboriculteurs sont confrontés à une hausse sans précédent par son ampleur et sa rapidité des coûts de production. L'augmentation du prix de l'électricité de l'eau des emballages ont conduit à une hausse de 8% du prix de vente des produits. Dans le même temps des pommes extra-hexagonales sont proposés à la vente avec un prix inférieur de 7%, en concurrence avec des fruits défiant les normes sanitaires respectés par nos arboriculteurs prise en étau, les arboriculteurs en arrivent à arracher des Pommiers afin de ne pas vendre à perte, leur production. Les plus petites exploitations n'arrive plus à assurer un niveau de revenu décent pour leur agriculteurs ce qui n'est pas acceptable. Madame la Ministre, voilà une partie de notre Patrimoine alimentaire qui est aujourd'hui menacée. Alors que l'approvisionnement de nos pommes s'avère de plus en plus dépendante de prix cassés et de normes sanitaires dégradées. Commun Madame la Ministre. Entendez-vous nous aider à préserver la production de grande qualité des arboriculteurs deux autres provinces. Je vous remercie. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, le Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire à échanger avec les professionnels arboricole sur les difficultés de la filière lors de son déplacement à Angers au Salon international des techniques de production végétale Première éléments le prix du kilo de pomme, c'est tout l'enjeu de la loi Egalim de qui ne couvre pas les fruits et légumes à leur demande, c'est un regret, il faut sans doute se poser la question et y travailler car pour protéger la rémunération des agriculteurs. Il nous faut des contrats conclus dans le cadre de cette loi le bon prix c'est celui qui permet de rémunérer le producteur 2ème. Sujet de préoccupation, le retrait des produits phytosanitaires et difficultés liées à la protection des végétaux. Il nous faut penser des transitions ambitieuse et soutenables sur le territoire européen afin qu'elles ne soient pas pénalisantes pour les producteurs français tout en s'assurant de la nécessaire réduction des usages. C'est une nécessité par exemple sur les néo-Cottineau hein ou pour le foie se mettent pour la filière cerise. La France s'assure que nous ayons une action européenne coordonnée en la matière et va déclencher une clause de sauvegarde afin d'éviter toute distorsion de concurrence. C'est cette logique de la réciprocité des normes et des clauses miroirs que nous devons défendre dans les accords commerciaux en parallèle de notre ambition partagée de transition écologique. Enfin il faut anticiper en développant la recherche d'alternatives afin de ne pas laisser la filière sans solution technique, c'est aussi un des enjeux des renouvellements de vergers, actuellement de 4,2% avec de nouvelles variétés plus résistantes monsieur adaptée au climat. C'est tout l'enjeu de la planification écologique. Le plan de souveraineté, fruits et légumes en cours de finalisation, qui sera présenté au salon de l'agriculture intégrera ses dimensions et les enjeux d'innovation au coeur de la 3e révolution agricole nous conduirons ce chantier visant à inverser à horizon 2030, la tendance baissière de notre souveraineté sur ces filières dans cette logique de transition et de planification. Merci monsieur Roux, vous avez 19 secondes. Merci madame la présidente. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Et vous savez c'est un, un jeune important au niveau des agriculteurs et surtout les arboriculteurs par rapport à cette concurrence et que nous avons et aujourd'hui malheureusement ils sont tombés obligé d'arracher des pommiers par rapport pour essayer d'équilibrer leur budget. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Annie Le Houerou. Merci. Si madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, ma question porte sur les soutiens urgent à apporter à la filière porcine biologique qui s'effondre en Bretagne. La filière porcine s'est organisé pour répondre à une demande croissante en porc biologique. Or depuis le second semestre 2021 la consommation de la viande de porc La filière porcine bio et de ce fait, en situation de surproduction qui l'a contraint à baisser ses prix en s'alignant sur ceux des ports conventionnelle ce déclassement ne permet plus aux producteurs biologiques de couvrir leurs coûts de production. L'augmentation du prix des matières premières, de l'alimentation et de l'énergie, conjuguée à la l'amortissement des investissements qui ont été nécessaires à la conversion en agriculture biologique notamment l'adaptation des bâtiments mais les producteurs en très grande difficulté. L'avenir de la filière porcine biologique et donc en danger, alors même que l'objectif fixé par le plan de développement de la filière porcine française, de passer de 0 5 % à 5% de production porcine biologique est loin d'être atteint en France en 2021, seul 1,45% des porcs abattus était biologique. La loi du 30 octobre 2018 Egalim complétée par la loi climat dite de climat et résilience prévoit au moins 50% de produits de qualité, durable, dont au moins 20% de produits biologiques dans la restauration collective, nous en sommes très loin dans nos écoles, collèges, lycées, hôpitaux, établissements médico-sociaux. Le seul respect de cette loi permettrait d'éviter la situation de surproduction que je viens de vous évoquez et garantirait la pérennité de la filière porcine bio en Bretagne et en France l'agriculture biologique a un impact positif sur la santé, le climat, la biodiversité et les diverses pollutions elle répond assurément aux enjeux agricoles sociétaux actuels et futurs, madame la Ministre, que prévoit le gouvernement pour venir en aide d'urgence aux producteurs devant de viande bio qui se trouve dans un désarroi total sans soutien d'urgence et producteurs de Plouisy de Pleo de Plélo et d'ailleurs court à la catastrophe mais avec des dégâts humains que l'on sait. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, madame la sénatrice m'interroger sur la situation de la filière porcine biologique en Bretagne et sur le territoire national. Rien n'indique que l'atteinte de l'objectif de 20% de produits bio servis en restauration collective augmenterait de façon significative les achats de porc bio en effet les restaurants collectifs non pas en effet l'obligation de servir de la viande de porc bio et peuvent retenir d'autres productions sans label biologique et même d'autres labels pour le port voir aucun Label la difficulté de la filière porc bio est avant tout d'arriver à mieux valoriser ses produits et notamment toute la carcasse de porc à ce jour dans la majorité des cas, seule une partie de la carcasse et valorisées en agriculture biologique notamment les jambons le reste intègre les circuits conventionnels 2ème difficulté produire du porc bio nécessite des bâtiments d'élevage et une organisation de production qui génère des surcoûts importants. Cela rend impossible de déclasser transitoirement les viandes en conventionnel, comme peuvent se le permettre d'autres filières car les pertes financières sont vite intenable. Le ministre a annoncé aux assises de la bio. Le 6 décembre 2022, un projet de structuration de la filière porc bio et le travail a été engagée avec l'Agence Bio et le représentant de la filière un abondement du Fonds Avenir Bio de 2 millions d'euros supplémentaires à destination des filières bio les plus impactés dont la filière porc bio, une campagne de communication à destination du grand public doté de 750.000 euros pour augmenter la demande réitération de la campagne. Réflexe de 2022. Une campagne de communication lancée en 2023 grâce au financement du programme de promotion européen qui doit permettre de stimuler la consommation en restauration commerciale. Enfin, le ministère a ouvert la possibilité aux régions qui le souhaitent de mobiliser les reliquats du Feder 2014 2022 pour mettre en place en 2023 une aide au maintien à l'agriculture biologique. La région Bretagne. La mise en place par ailleurs le futur programme Ambition bio sera l'occasion de construire avec les filières et les acteurs du bio, une véritable stratégie renouvelée d'accompagnement et de structuration de ces filières de qualité tenant compte des résultats des études prospectives en cours qui d'ailleurs seront l'occasion de mieux équilibrer l'offre et la demande. La parole est à monsieur le président Jean-François Longeot. Merci madame la présidente, madame la ministre. Chaque année la conchyliculture est touché par des épidémies de norovirus qui sont en grande partie causée par les problèmes persistants liés au traitement des eaux usées dans les zones littorales. À la faveur des épidémies hivernales sévissant chez les être s'humains certains virus deviennent présent en grande quantité dans les eaux usées et il apparaît qu'une partie d'entre eux ne parvient pas à être détruite lors des phases de traitement. Ainsi nous assistons régulièrement à des épidémies de contamination des huîtres du fait des nos norovirus responsable du virus de la gastro-entérite, quelles mesures concrètes, le gouvernement compte-t-il prendre pour aborder ces problèmes de manière efficace et garantir la sécurité sanitaire des consommateurs de produits de la mer. Les ostréiculteurs se retrouve touchée par les restrictions de production ne sont aucunement responsables de la situation mais en paix. Pourtant le prix fort. Comment le gouvernement peut-il mettre en place un mécanisme pérenne qui permette de soutenir nos ostréiculteurs face à ces aléas. Lors d'une question d'actualité posée en 2020, il y aura un épisode de crise de la conchyliculture. Le gouvernement s'était engagé à améliorer le contrôle du traitement des eaux usées en adressant des instructions aux préfets pour renforcer les contrôles sur les 1 pendages dans les zones concernées. Pourriez-vous Madame la Ministre nous informer de l'avancement de cette stratégie et de l'impact qu'elle a eu sur la situation actuelle des épidémies de norovirus la conchyliculture, je vous remercie. Merci la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur. D'abord je prie de vouloir excuser l'absence de secrétaire chargé de la mer à 20 Berville qui n'a pu être présent ce matin vous nous interrogez sur l'enjeu de la conchyliculture et la normande, que je suis ne peut être qu'attentive à ces questions. Un fléau qui est bien identifié comme vous l'expliquait très justement les cultures conchylicole ont été touchés de plein fouet cet hiver par les contamination au norovirus en pleine période de fêtes de fin d'année. Elles ont entraîné d'importants préjudices pour la filière. Le gouvernement suit ce sujet avec attention et travaille à des solutions de court et de moyen terme. Des actions sur la qualité du milieu. Parmi elles, la mise en conformité des systèmes d'assainissement avec l'augmentation des populations côtières et l'évolution de la réglementation environnementale. Mais ce sont des chantiers longs et complexes. Face à l'urgence de la situation, les ministres en charge de l'écologie de l'agriculture et de la mère travaille avec les préfets pour lancer rapidement les travaux de mise en conformité pour les zones à usage sensibles comme celles destinées à la conchyliculture en état des lieux sera demandé pour lister les chantiers prioritaires valoriser les bonnes pratiques et identifier les blocages un plan d'action est un soutien financier. Le gouvernement va également travailler sur un plan d'action avec les collectivités concernées qui sera complémentaire à ces travaux. Enfin un accompagnement financier pour être proposées aux conchyliculteurs notamment via le fonds européen pour les Affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture ces aides à l'investissement pourront financer des bassins de mise à l'abri ou de purification des systèmes d'alerte des projets portés par les régions ou encore la constitution d'un système d'assurance pour laquelle l'État est prêt à accompagner la profession.

Mais c'est aussi un sujet d'avenir pour les ostréiculteurs. Et je pense qu'au-delà des accompagnements qu'on pourrait mettre en place que le gouvernement pourrait mettre en place. Je crois qu'il est temps que pour l'ensemble de traitement de nos stations d'épuration, on est des, des techniciens qui puisse adapter nos modes de traitement à nos modes de vie actuel, merci. Merci. Je remercie même la ministre Firmin Le Bodo, pour la gestion du temps également parfaite comme son collègue précédent. Merci. La parole est à madame Véronique Guillotin. Merci madame la présidente, madame la ministre, vous connaissez certainement la situation de l'accès aux soins dans notre pays et j'entrerai pas dans les détails, car tout le monde peut malheureusement expérimenter au quotidien les difficultés je vous parlerai en fait d'Europe et de ceux qui la vivent au quotidien en habitant dans une zone frontalière, c'est le cas dans le nord de la Meurthe-et-Moselle et le nord mosellan et notamment à la frontière avec le Luxembourg qui attire chaque année de plus en plus de travailleurs sans-12.000 Français y travaillent en 2021, il travaillait dont plus de 30.000 qui vivent sur cette bordure transfrontalière. Pour eux et pour tous ceux qui habitent dans cette zone. La frontière n'est qu'une réalité administrative tant les échanges et les déplacements entre les 2 pays sont fréquents, malheureusement l'administration précisément vient compliquer leur quotidien alors que l'accès aux soins devient de plus en plus compliqué. Du côté français, y compris du fait de l'aspiration massive des professionnels de santé au au Luxembourg de nombreux frontaliers voudrait voir certains verrous administratifs levé ce qui demande à l'assurance maladie de de valider le remboursement d'une consultation Luxembourg se voient souvent opposer l'absence de pertinence de soins souhaité lorsqu'il n'abandonne pas eux-. Mêmes les démarches du fait des complications administratives trop longue et trop complexe pour éviter cela dans certaines zones frontalières françaises, belges et allemandes les populations, établissements de soins et professionnels de santé ont émis le souhait de mettre en oeuvre des dispositifs de simplification administrative et financière, en matière d'accès aux soins à l'étranger. Il s'agit de ce que l'on appelle des zone d'organiser Dax zone organisée d'accès aux soins transfrontaliers. Mais aucune n'a vu le jour entre la France et le Luxembourg, nous travaillons déjà sur de nombreux projets communs au sein du groupement européen de coopération territoriale territoriale le GE c'était la zone ouest à Paris donc pour nous, plus particulièrement une solution pertinente et souhaitable, je souhaiterais savoir si le gouvernement entend se saisir de ce sujet qui nécessitent une intervention des 2 États. la parole est à madame Chrysoula Zacharopoulou Secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux et bonjour, madame la Ministre bonjour, madame la présidente. Madame la sénatrice Véronique Guillotin. Je vous prie tout d'abord d'excuser Madame la secrétaire d'État chargé de l'Europe qui m'a chargé de vous répondre. Comme vous savez, la pandémie a renforcé les difficultés de certains de nos concitoyens en matière d'accès aux soins, tout en mettant en lumière la forte sur qui pesait déjà journaux le système de santé. Pour cette raison, la santé et avec les transports. La première des attentes des noms citoyens vis-à-vis de la coopération frontalière le développement d'une offre un mutualiser aux frontières est une façon efficiente. Améliorer l'accès aux soins à 100 pillant sur des ressources médicales déjà existantes et en simplifiant les démarches administratives pour nos concitoyens. C'est bien l'objectif, comme vous l'avez dit des concepts, des zones organisée d'accès aux soins. Transfrontalière. C'est là, par exemple, été développé dans les yeux le District. Moselle à travers la confession de Mozart et plus récemment par la Constitution expert. L'ARS Occitanie aussi piloter un projet d'établissement de santé binational entre la France et l'Espagne. Et combien toutefois de noter que le déploiement de tels mécanismes est complexe, elle n'apporte pour l'instant qui ne réponse partielle aux difficultés des des noms qu'citoyens. L'implication des des systèmes de santé nationaux appliquent en effet il ne préparation et de mise en oeuvre important qui mobilise dénombré moyen jouera ensemble des sujets fondamentaux ne réflexion n'a été entamé entre les services des ministères de la Santé français et celui des Luxembourg sur la mise en place d'un tel dispositif entre nos 2 pays, je vous remercie. Merci même Guillotin, il voudrait se disent 12 secondes. Je vais les prendre. En tout cas j'ai entendu que le le sujet avancer, je pense que si ça existe si c'est possible entre la France et la Belgique. Ça doit être possible entre la France et Luxembourg. Je pense que c'est une vraie difficulté en tout cas sur le territoire français. Les 2 pays serait gagnant gagnant. Je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui accélérer et arrivé à nous faire avoir un petit peu d'horizon un peu plus clair en tout cas entière de m'accès aux soins et cet OS pourrait y participer. Madame la Ministre. Collègues. La parole est à monsieur Pierre Ouzoulias. Merci madame la présidente. Madame la miss mais mes chers collègues. Pendant la guerre des 40 jours que l'Azerbaïdjan a livré contre la petite république. D'tsar. Puis de nouveau en septembre 2022. L'armée azérie s'est livrée à des exactions contre les militaires en en violation du droit international, mais aussi contre contre les civils. Ma première question est, est simple. Quelles sont les, les initiatives que va prendre la France pour faire reconnaître les crimes de guerre par les instances internationales. Depuis le le 12 décembre. 2022, c'est-à-dire depuis 2 mois. L'Azerbaïdjan a mis en oeuvre un un blocus militaire de la République d'tsar. 120.000 Arméniens sont privés de tout. Et l'Azerbaïdjan ne leur laisse le choix qu'entre fuir ou bien périr. La France et l'Europe ont des moyens de pression sur l'Azerbaïdjan. Pourquoi ne les utilise-t-elle pas. En 1939, la France a abandonné à la Turquie le Sandjak d'Alexandrette condamnant ainsi à l'exil. 5 50.000 Arméniens allons-nous une nouvelle fois abandonné la République d'tsar. Merci, madame la Ministre. la parole est à madame Chrysoula Zacharopoulou Secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Monsieur le sénateur. Oh Julia. Lors de l'offensive hein azerbaïdjanaise de 13 et 14 septembre 2022. La France a immédiatement dénoncé la violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie et appelé. Au retour des forces azerbaïdjanaises à l'air précision initiale des plus et comme elle a fait des piles déclenchement de la guerre du rock à Rabat en 2020 la France a dit qu'est les crimes de guerre devait être jugeait l'air other puni. La lutte contre Hippolyte est essentielle pour offrir enfin aux populations de la région Île perspectives de paix. La réunion organisée par le président de la République à Prague le 6 octobre 2022 a présence de Messier Nikol Pachinian Ilham Aliev, Charles Michel a permis d'obtenir un accord pour l'envoi d'une mission de la baisse décès civils qui se déployait pour des mois un territoire arménien. Elle a contribué à faire baisser la tension. Sur le terrain et le nombre des accidents significatifs a diminué après ses bons résultats nos efforts ont concouru assez qu'17 décide le 23 janvier 2023. Le déploiement d'une mission d'un territoire arménien pour 2 ans cette fois-ci, la France et contribuer la par la voie des gendarmes. La diplomatie française est mobilisée au plus haut niveau pour permettre une paix juste et durable dans le Caucase du Sud au bénéfice des populations. Cette mobilisation qui est la nôtre depuis plus de 30 ans poursuit aujourd'hui avec la même détermination, comme le montrait encore la semaine dernière les échanges entre le président de la République et ses homologues arméniens et azerbaïdjanais azerbaïdjanais. Je rappelle que la France n'apporte pas des casses a. Nous soutenons les efforts de la Commission européenne pour diversifier les approvisionnements énergétiques de l'Europe et de réduire notre dépendance au gaz russe

Madame. La Ministre. J'aurais aimé que la France reconnaisse la violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie, mais aussi de la république d'Artsakh. Est-ce que c'est la République tartare qui a été attaqué attaqué par. Par l'Azerbaïdjan je je pense qu'aujourd'hui la seule solution pour sauver ses 120.000 Arméniens de la République d'art. C'est une reconnaissance officielle par la France de la république d'Artsakh comme le Sénat. Vous l'a demandé à une très très large majorité. Vous m'avez répondu, mais vous n'avez dit aucun mot sur le blocage en cours de la république. D'Artsakh. Les gens manquent de tout. ils n'ont plus de nourriture, il y a des tickets de rationnement. Il y a plus de médicaments, il n'y a plus rien donc il faut agir maintenant. Merci ma président. Merci la parole est à monsieur Gilbert Roger. Madame la présidente, madame la Ministre. Avec la crise énergétique. Que la France et l'Europe connaissent le gouvernement a demandé aux Français. Une certaine sobriété énergétique, les dirigeants d'EDF et d'Engie en particulier souhaite que nos concitoyens et l'utilisation des appareils électroménagers. Pour éviter la surcharge. Du réseau électrique. Ces derniers suggèrent de déclencher les équipements à partir de 22h. Or les horaires 10h les horaires 10h creuses en tarif bleu sont actuellement différents selon les abonnements mais majoritairement. Compris entre 23h 36 très précisément et 7h 36. Aussi, je souhaiterais savoir quelles mesures pourraient être prises par le gouvernement pour uniformiser les abonnements élargir les horaires des heures creuses de nuit entre 22h 30 et 7h 30 et avec le décret autorisant les fournisseurs d'électricité à suspendre la tranche creuse entre 12h et 14h pour certains abonnements. Et via Linky. Cette proposition s'insérer dans la communication cohérente du gouvernement, je vous remercie. Merci la parole est à madame crise ou la saga Zacharopoulou Secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Mais si elle la Chaîne Inter Gilbert Roger, je vais vous répond au nom des des mon collègue Agnès Pannier Runacher ministre de la transfusion. Qui vous prie de bien vouloir excuser son absence. Les heures creuses des options Air pleines heures creuses sont aujourd'hui dans les plages de 12h à 17h et de 20h à 8h.

a conduit le gouvernement à demander aux gestionnaires des réseaux des procéder à la désactivation partielle pour l'hiver 2022 du démarrage des ballons d'eau chaude sur cette plage horaire sans accident sous la facture d'électricité, est-ce un accident sur le jazz de l'eau chaude qui stockent par nature la salaire c'est la permis des décalé pendant la nuit, une consommation équivalent à la production des plus de 2 réacteurs nucléaires, renforçant ainsi la résilience des notre système électrique. La ministre de la de rescision énergétique souhaite développer encore plus les signaux tarifaires. À l'instar des offres Tempo qu'ils en ont augmenté fortement, à 2000, vendait sous son impulsion, je vous confirme qu'il n'évolution désert. Également un cours d'expertise. Merci monsieur Roger vous avez 38 secondes. Je vais pas utiliser les 38 secondes mais. J'espère que, très rapidement, on pourra arriver à l'idée que de 22h à 7h 30 et non pas 23h 36. Les heures creuses s'établissent. Il y a pas besoin d'avoir une commission très longue pour décider de cela donc. Attendons. Rapidement une décision. Merci. Merci la parole est à monsieur Philippe mouiller. Merci madame la présidente, madame la ministre. Ma question s'adresse à Madame, la ministre de la transition énergétique et porte sur les conséquences financières de l'envolée de la volatilité des prix de gros de l'électricité pour les acheteurs obligé. un moment à l'article L 121 6 du code de l'énergie, ceux-ci sont tenus de rembourser à l'État le différentiel entre la valorisation qu'ils font des production d'énergies renouvelables et le prix d'achat garanti auquel ils les ont acquises. Toutefois, en l'état aucun texte n'encadre les modalités dans lesquelles évaluer ses recettes et effectuer leurs renversement au profit de l'État. En effet, c'est l'article L 121 6 du code de l'énergie prévoit bien le reversement des recettes induites par les obligations de service public en particulier pour les acheteurs obligé la loi n'habite la à intervenir que lorsque les obligations de service donne lieu à une compensation par l'État des charges qu'elles induisent. Pour les opérateurs. Cette situation inédite n'avait pas été anticipé par le législateur ni à pourrir surpris par le pouvoir réglementaire. Ainsi les articles R 121 22 et suivants du code de l'énergie n'encadre que des opérations de compensation par l'État des charges induites par les obligations de service public et non celles liées au reversements lorsque les dites obligations de lieu à des recettes pour les opérateurs concernés. C'est dans ce contexte que la créa délibéré le 3 novembre dernier afin de réévaluer les recettes désigné par l'Autorité de régulation. Et donc ses recettes ayant déjà fait l'objet d'une délibération le 13 juillet 2022. Cette nouvelle évaluation qui se font notamment sur des réalités de marché de gros, très évolutive et de nature à mettre en grande difficulté. Les acheteurs obligé et parmi eux les entreprises locales de distribution. En effet, les charges de trésorerie qui résulte de l'écart destination basé sur la délibération de novembre les pousserait notamment à des cessions de paiement dès dès dès Ainsi est-il envisagé d'établir un cadre légal et réglementaire plus sécurisant pour les acheteurs obligé et plus particulièrement pour les ALD. Je vous remercie pour votre réponse pour cette questions techniques. Merci. La parole est à madame Chrysoula 5 Poulloux secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie.

Comme voulait rappeler la situation actuelle conduit à une. Contribution de positive des énergies renouvelables aux finances publiques. La réévaluation exceptionnelle des charges de service public en novembre 2022 a en effet conduit à un ajustement des nouveaux reversement dans un contexte où les prix des marchés en dépit baissait. Pourra pallier à ces sujets d'une part, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé aux opérateurs son engagement de réviser ses évaluations des charges pour l'année 2023 faire à l'occasion des sa délibération dès juillet 2023, ce qui permettra une arrêt qui brasse des de reversement. D'autre part, les services de l'État proposeront. aux acteurs concernés et notamment étais prise local de distribution des solutions transitoires, y compris conventionnelle afin de pouvoir éviter les cas où un stress de trésorerie serait insupportable au première semestre 2023. quarts de versements contrainte on essaiera initié si un doute persiste sur son montant. Je vous remercie. Merci la parole est à madame Brigitte de. Madame la présidente, madame la Ministre, le 11 février 2022, l'État a annoncé la construction d'une nouvelle cité judiciaire à Marseille à l'horizon 2028. Elle occupera 40.000 m2 de locaux et réunira 600 magistrats et fonctionnaires. Dotés enfin la 2ème ville de France, d'un site unique où se regrouperont toutes ses activités judiciaires, permettra de mettre fin à l'éclatement géographique des juridictions marseillaise qui ne facilite pas le travail de l'ensemble des acteurs de la justice. En cela, l'initiative de l'État va dans le bon sens et il convient de le souligner. Cependant à seulement 5 ans de la date annoncée par la fin de sa construction. La localisation de cette future cité judiciaire n'est toujours pas connue. 3 sites sont envisagés le centre-ville de Marseille qui semble être l'option privilégiée mais aussi les sites d'euro Méditerranée de et de La Capelette. L'absence à ce jour d'une feuille de route expliquant la méthode retenue tant pour choisir le futur site ainsi que le choix de l'architecture intérieure pose question pour faire aboutir ce projet, il sera nécessaire de consulter tous les acteurs du monde judiciaire marseillais et notamment les avocats qui, par leur voix de leur bâtonnier ainsi que de l'Union des jeunes avocats de Marseille font part de leur vive inquiétude sur l'emplacement du site à plus de 99% selon un sondage en effet étant installé dans des cabinets très souvent situés à proximité des tribunaux actuels, ils seront les premiers impactés par la nouvelle localisation des juridictions marseillaise. Or aucune consultation de nature n'a pour le moment été annoncé Madame la Ministre, ne pensez-vous pas que la participation des avocats au sein du conseil d'administration de la pige, agence publique pour l'immobilier judiciaire seraient souhaitables, ceci afin de pérenniser le dialogue sur l'architecture et l'organisation des palais de justice. Par ailleurs, l'État doit expliquer quel sera le processus de concertation envisagée pour aboutir à la décision définitive en effet l'État étant le principal acteur et promoteur de ce site ne devrait-il pas indiqué vers quel emplacement va actuellement sa préférence pour la construction de la cité judiciaire de Marseille. Je vous remercie. Si la parole est à madame Chrysoula Zacharopoulou Secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. je vais vous répondre au nom de mon collègue Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice, ce que vous prie de bien vouloir excuser sur l'absence qu'un retenus par des autres obligations. Les ministres, annoncé en février dernier, les projets de construction de la cité judiciaire de Marseille, afin de regrouper les juridictions marseillaise au sein d'une même bâtiment fonctionnel et adapté à la justice du XXIe siècle. Les réflexions pour définir les meilleurs sites se poursuivent antenne seulement avec les services en charge de la nettement au bas. D'une part et en concertation permanente avec les élus locaux, d'autre part l'ampleur des gens j'ai liés à ces projets nécessitent que le gouvernement prenne prenne le temps de la réflexion et surtout de la concertation. Les garde des Sceaux et d'ailleurs un lien permanent avec les maires des Marseillais est la présidente de la métropole à ce stade les nombreuses contraintes fonctionnelles des sites actuels interroge quand la possibilité d'offrir aux juridictions marseillaise à la fin une cité judiciaire. Et un outil de travail et fonctionnelles sécurisées et conforme aux orientations du gouvernement en matière de développement durable. Par contraste, l'option d'une construction neuve et fonctionnelle. Permettrait à la fois de regrouper l'assemble des juridictions dans un seul bâtiment moderne et performant d'impôts énergétique et c'est dans un calendrier beaucoup plus resserré. C'est sur cette base, madame la sénatrice qu'elle. Le ministre de la justice souhaite poursuivre la concertation avec l'salle des parties concernées dont les magistrats, greffiers et avocats dans l'objectif d'apporter très rapidement ah Meyer, service public de la justice à l'auteur des attends des Marseillais. Je vous remercie. Merci la parole est à madame Marie-Arlette Carlotti. Merci madame la présidente, madame la ministre, il y a 10 ans, 3 femmes 3 militantes de la cause kurde ont été assassinés en plein Paris. Sakine Fida Leila ont été les premières à scander ce slogan qui est désormais le symbole de courage des femmes iraniennes, femme, vie, liberté, mais justice n'a pu être rendu. Le principal suspect a toujours nié les faits et il est mort en décembre 2016 quelques mois moi avant son procès. Depuis 10 ans. Les familles des 3 victimes attendent la vérité une vérité qu'on leur cache et qu'on nous cache puisque les autorités françaises refusent toujours la déclassification des documents détenus par les services secrets français. La juge d'instruction antiterroriste qui a renvoyé aux assises Omer Güney pour ce triple assassinat avait pourtant pointé des accointances du suspect avec les services secrets turcs mais la commission consultative sur le secret défense n'a autorisé la divulgation que de 36. Document et le suspect était bel et bien écouté par les services secrets français, mais le contenu des conversations n'a pas pu être déclassé. L'enquête judiciaire n'est donc pas terminée. Les avocats des victimes ont saisi le parquet afin de reprendre l'enquête pour que soient identifiés les commanditaires. Nous ne pouvons accepter Madame la Ministre que de liquidation physique soit perpétrés sur le sol français. Alors que les 250.000 Kurdes qui vivent en France ont été extrêmement marquée par ces assassinats. 10 ans après un nouvel événement sanglant est venu recours réouvrir leurs blessures. La communauté kurde a été de nouveau touché à Paris ce 23 décembre. Des morts encore des morts. Désormais à la peur, peur de vivre dans le pays où elle a pourtant trouvé refuge le pays des droits de l'homme, la France est le pays des lumières, madame la Ministre, le gouvernement aura-t-il désormais le courage de lever le secret défense contre sur tous les éléments de ce dossier. Merci de votre réponse. Merci la parole est à madame Chrysoula Zacharopoulou Secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la sénatrice Marie-Arlette Carlotti, je vais vous répondre au long de mon collègue Sébastien Lecornu, ministre des armées qui vous prie de bien vouloir excuser son absence la 9 janvier 2013, 3 en cours on était assassiné dans le dixième arrondissement de Paris près de 10 ans avant le drame qui a de nouveau endeuillé ces quartiers en décembre dernier, comme vous l'avez rappelé dans votre question, nous avons une pensée pour ses victimes et leurs familles. Des pays 2013. Le ministère des Armées a été sollicité afin de transmettre à la justice des documents relatifs à ces crimes. Ainsi en 2015 le ministère des Armées à déclassifier ces documents après avoir saisi la commission des secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative Independent qui a été créé pour donner un avis indépendante sur les des classifications, la communication d'informations. Ayant fait l'objet d'une classification, cette commission est constituée d'un même des conseillers d'État des magistrats de la Cour de cassation des magistrats de la Cour des comptes d'un député hein c'est Inter le ministère des Armées indique qu'ils ne détiennent aujourd'hui plus de documents pouvant concourir à la manifestation de la vérité, je vous remercie. Merci beaucoup madame Carlotti, vous avez 12 12 secondes. Hé bien je voulais dire que le 21 mars, ce sera le nouvel an kurde et pour ce jour-là ce jour-là. Nous espérons vraiment cette fois une réponse positive. Merci. Merci beaucoup et merci madame la ministre a bonne gestion de votre temps, ce qui donne beaucoup de pression pour votre collègue qui arrivent derrière parce que nous n'avons eu que des bons élèves ce matin. C'est pour le temps de parole. Voilà. Bonjour monsieur le Ministre. La parole est à monsieur Didier Mandelli. merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question concerne le raccordement en fibre optique des villes des sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon en Vendée situé en zone d'appel à manifestation. D'intentions d'investissement hein plaise au On a fait le raccordement en fibre a pris un retard important pour ces 2 villes environ un quart des foyers de ces 2 agglomérations ne sont pas encore accordé les pénalisant dans leur attractivité. Ainsi, seuls 77% des locaux sont raccordables en 2022 par rapport à la base réelle de logement et non pas ce qui. À l'origine aux sables d'Olonne agglomération et seuls 70,7% des 59.701 locaux sur le territoire de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Ce qui est loin des engagements d'un raccordement à 100% pour 2020, nous sommes en 2023. Face à cette situation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'Arcep a mis en demeure Orange fin décembre 2022 pour ses retards. Il a également ouvert une procédure d'éventuelles sanctions. Pour les manquements dans ses engagements, j'ai interrogé la présidente de l'Arcep. La semaine dernière sur ce sujet en commission, elle s'est dite plutôt favorables à la reprise en main du déploiement de la fibre par les collectivités, si les opérateurs venait à manquer à leurs engagements. Je souhaiterais donc connaître les actions envisagées par le gouvernement et sa position pour répondre à ces situations, notamment sur l'annulation des contrats avec les opérateurs qui ne respectent pas les contrats passés avec les collectivités. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. d'un d'un arrêté qui acceptait les engagements proposés par Orange, dans le cadre de l'article L. 33 13 du code des postes et des communications électroniques avec des échéances en 2020, vous l'avez dit et 2022. Le gouvernement est pleinement conscient des efforts de l'ensemble des acteurs concernés par le déploiement et la réalisation du France très haute du plan pardon France très haut débit. Donc, il faut reconnaître qu'il est relativement ambitieux et dans l'ensemble plutôt assez bien livrer livrer si je puis dire notamment quand on se compare à nos, à nos partenaires européens. Cet enjeu a été particulièrement prégnant du fait de la crise sanitaire qui aurait pu ralentir durablement les déploiements et il faut le reconnaître, d'un certain nombre d'enjeux d'efficacité opérationnelle de sous-traitants d'Orange. Congé d'ailleurs la charge. De traiter les enjeux financiers qui m'occupe souvent à Bercy. Vous l'avez dit, au regard des données chiffrées issu de l'Observatoire de l'autorité de régulation, il est apparu que dans certains départements dont le vôtre. Les objectifs ne sont pas au niveau. C'est la raison pour laquelle l'Arcep. Vous l'avez dit, sur demande du gouvernement a ouvert une procédure prévue à l'article 36 11, aboutissant à une mise en demeure. Cette décision, vous le savez aussi a été attaqué par l'opérateur devant le Conseil d'État qui instruit actuellement le dossier. Nous sommes donc en attente de la décision du Conseil d'État suite à cette procédure. vous le savez, soyez assuré que le gouvernement est entièrement mobilisé pour rendre effectives les promesses présidentielles. La France s'est fixé un objectif ambitieux, celui de la généralisation des réseaux en fibre optique, horizon 2025 et Ford la conviction que la diffusion des réseaux en fibre est un levier d'attractivité des territoires. Le gouvernement se mobilise pour éviter que le numérique ne soit sur de fractures au sein de votre pays, vous avez cité des chiffres pardon pour les deux communes importantes de votre département d'autre chiffre malheureusement sont même en deçà et donc nous devons vraiment profité je dirais des deux 3 années qui viennent pour accélérer le mouvement malgré les défis que vous mentionnez. Nous avons monsieur le sénateur, tous ces tous tous ces tout hein pardon à coeur de trouver des solutions rapides et efficaces pour que les citoyens de département puissent bénéficier d'un accès à la fibre, l'une des pistes de réflexion peut également être la reprise en main des engagements de l'opérateur par des acteurs économiques locaux afin de mener à terme l'installation du très haut débit dans les Territoires. Merci, monsieur le Ministre, n'oubliez pas. Le. Monsieur Mandelli, vous avez 37 secondes. Oui madame la présidence ce sera plus ce qu'il n'en faut. Monsieur le Ministre. Moi je souhaite effectivement que nous puissions travailler sur la dernière hypothèse que vous avez évoquées, c'est-à-dire la possibilité pour les collectivités que local en lien avec les les réseaux d'initiative publique notamment dans le département de la Vendée de reprendre à leur compte l'ensemble des des opérations qui ne sont pas réalisées par l'opérateur historique. Merci la parole est à monsieur François Calvet. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur les conséquences de la hausse des prix de l'électricité. Pour notre Patrimoine religieux. En effet, si le gouvernement a déployé, d'une part un tarif un bouclier tarifaire permettant de plafonner la hausse du prix de l'électricité pour les particuliers et les petites entreprises et d'autre part, un dispositif de minoration des tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour les autres entreprises. Il a, il apparaît que ce dispositif qui concernent uniquement les tarifs réglementés dit bleu ne permet pas à tous de supporter la hausse du prix de l'électricité, la hausse des tarifs de l'énergie a également une incidence sur les édifices religieux à cet effet les gestionnaires des diocèses s'alarme face à l'augmentation de la facture énergétique. Ils ne peuvent pas faire face à ces nouveaux coups ainsi pour réduire à la fin, la facture énergétique souvent astronomiques dans les édifices au volume abyssaux des prête d'hésitent plus à tout éteindre et appelle les fidèles à se vêtir chaudement pour les cérémonies. Si la loi du 9 décembre 1905 pause à un son article 2, le principe de l'interdiction de subventionner les cultes. Il faut rappeler que le législateur a autorisé dans le texte voté en 1905 puis ultérieurement des exceptions à cette interdiction, puisque l'entretien des édifices religieux et confiée aux communes depuis 1907, la réalité est donc bien plus complexe. Aussi, sites. Cette situation, je vous demande si vous envisagez d'éteindre le dispositif d'aide. En la matière aux bâtiments religieux et les salles annexes utilisé pour l'enseignement religieux. Si la parole est à monsieur Roland Lescure Ministre délégué chargé de l'industrie. Si Madame le président. La présidente. Merci monsieur le sénateur Calvet pour votre question importante. Qui me permet de rappeler même si je ne vais pas les détails, vous l'avez dit, le nombre d'aides importants qui ont été mises en place par le gouvernement pour accompagner l'économie française et au fond la France et au fond la France dans son ensemble dans une situation difficile. La crise en Ukraine et la guerre en Ukraine d'ailleurs s'est traduit par une véritable crise énergétique une forte hausse des factures pour nos concitoyens. Elle a été très largement limité par le bouclier tarifaire voter dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et prolongé en 2023. Vous l'avez dit, des mesures spécifiques sur les TPE, les PME et les grandes entreprises, tout ça évidemment coûte beaucoup d'argent et ne permet pas malheureusement de couvrir tout le monde et notamment vous l'avez dit, les édifices religieux qui ne sont pas directement concernés. J'en profite quand même avant de répondre à votre question, pour appeler à nouveau les TPE et les PME à se signaler auprès de leur fournisseur d'électricité pour qu'il puisse bénéficier du dispositif d'aide. On a encore insuffisamment. d'entreprises éligibles. Aujourd'hui qui de fait font la demande, c'est quand même dommage de reconnaître que dans certains secteurs on n'y a pas droit et qu'on aimerait en avoir droit et que d'autres. On y a droit et qu'on ne fait pas appel donc c'est, c'est un message très important et je vous remercie monsieur le sénateur, de me permettre de le rappeler en ce qui concerne votre question. Je naïve 1000 de jeunes là limiterai pas pardon aux seuls édifices religieux à tous les édifices détenus par des associations cultuelles singulièrement les associations diocésaines ainsi qu'aux établissements de l'établissement catholique et d'autres lieux d'accueil du public dont beaucoup d'entre eux vous l'avez dit, ne sont pas couverts par les dispositifs, je peux vous dire que le gouvernement travaille encore à des mesures complémentaires les visant qui pourrait prendre deux formes. Hein. Évidemment et c'est l'enjeu majeur les appuyer dans la transition énergétique, de manière à ce que leur consommation d'énergie, baisse de manière durable. Mais aussi peut-être à court terme pour accompagner les gestionnaires de ces auditions. Ce que je peux vous le dire pour avoir échangé avec monsieur le ministre de l'Intérieur, pas plus tard que ce matin à ce sujet, il réunit l'instance de dialogue avec l'église catholique au mois de mars et il a prévu d'échanger avec leurs représentants pour évoquer les différentes solutions possibles et j'espère en trouver qui satisferont les acteurs merci. Merci monsieur Ministre Monsieur Calvez merci. La parole est à madame Christine Lavarde. Merci madame la présidente. Alors Monsieur le Ministre, je ne vais pas vous présenter les dark stores les Dark kitchens et les nuisances qui vont avec. Je suis sûr que ça vous connaissez, je vais aller droit au but et vous poser de question, quelle est la qualification juridique de ses locaux. Est-ce des entrepôts, des commerces ou des espaces de logistique urbaine telle que l'a qualifié le tribunal administratif de Paris en octobre 2022, justifiant cette définition car ces endroits permettrait de diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraisons dans Paris intra-muros ma 2ème question c'est, quid de la promesse de régulation du secteur au cours de l'été, les élus ont découvert par voie de presse. Un projet de texte réglementaire qui a entraîné un certain nombre, on va dire de propos plus ou moins vindicatif, le gouvernement a décidé de mettre rapidement. Une concertation qui s'est traduit par un communiqué de presse du 6 septembre qui a annoncé une réglementation rapide. Nous sommes près de 6 mois plus tard. Alors quelle est donc la cause de ce retard. Le commerce rapide c'est le commerce livré chez vous en quelques minutes les Dax que Store pardon comme les Dark kitchens sur la Pierre angulaire de cette nouvelle forme de commerce, il faut les distinguer des Drive puisque pour ces derniers. C'est le consommateur qui fait le déplacement. Exactement comme il le fait pour un magasin et vous l'avez dit, depuis quelques mois le modèle du Quick commerce fait débat. D'abord parce que son équilibre économique à loin d'être d'avoir été trouvé, il y avait 9 acteurs à Paris il y a un an, il n'y en a plus que trois aujourd'hui et tous les plans de développement ont été gelés. Il fait débat aussi et peut-être même surtout parce qu'il génère des nuisances de voisinage parce qu'il interroge aussi notre modèle de société et au-delà, notre modèle de consommation avec mon collègue Olivier Klein et les associations d'élus locaux. Nous nous sommes engagés à ce que ça faisait ses activités pardon, fasse l'objet d'une nouvelle régulation qui sera entérinée. Je vous l'annonce, dans un arrêté à paraître dans les prochains jours les dark stores seront intégrées dans la sous-destination d'urbanisme entrepôt pour répond de manière très concrète à vos questions. Qu'ils aient ou non un point de retrait. Alors qu'auparavant un point de retrait permettait de les considérer comme des commerces pour les Dark kitchens l'activité est tellement spécifique que nous allons créer une catégorie Haddock, ce qui a également été accepté par les élus. Nous entendons donc réglementer l'implantation des. D'accord et des Dark kitchens afin de permettre aux élus locaux de disposer d'outils pour les réguler, voire les interdire les PLU donne lieu à un zonage les élus peuvent autoriser autorisé sous conditions ou interdire les dark stores comme les Dark kitchens dans telle ou telle zone ces outils seront efficaces ne sont pas les seuls lorsqu'un appel Rather achète un commerce pour le transformer en dernière sort il devra solliciter l'accord préalable de la commune. Enfin et surtout, les mères dispose d'ores et déjà de pouvoir de police qui leur permettent de de réglementer. Les effets négatifs des dark stores, que ce soit en matière de regroupement de personnes devant un local d'interdiction de stationnement ou même de régulation. Vous l'avez dit-il, la circulation des 2 roues servant à la livraison. Nous sommes vigilants à ce que les élus soient dotés d'un arsenal complet pour encadrer la prolifération de ces nouveaux commerces et je le répète, un arrêté sera publié dans les prochains jours pour préciser tout cela. Merci, merci Monsieur le Ministre, même la vente, vous avez une minute. Oui alors dans quelques jours, j'aurais préféré que vous me disiez que l'arrêté été dans Solon parce que j'aurais été sûr comme ça que ça était vraiment imminents parce que les quelques jours c'est aussi un peu ce que vous aviez dit, pas vous mais vos collègues, le 6 septembre dans la conférence de presse. Ce dont je me réjouis, c'est qu'effectivement les deux catégories qui ont été choisies sont celles qui vont vraiment permettre de pouvoir limiter l'implantation de ces commerces qui sont vraiment des sources de nuisance. Et après vous m'avez reciter les pouvoirs qui sont à la main des maires pour essayer de réguler cette ses activités. Je suis au regret de vous dire que pour essayer de les expérimenter au quotidien, c'est assez compliqué et qu'on ne peut pas le faire sans un vrai partenariat aussi avec les entreprises qui utilisent notamment les Deliveroo les UberEats ou autres et que ça nécessite de mettre en place des solutions technologiques et donc il y a encore à faire, il faut le droit, mais il faut aussi la pratique et on avait besoin de cet arrêté donc merci et je vais être très vigilante sur les quelques jours. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur le président, Serge Babary. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Ma question porte sur la présence de substances dangereuses dans les fournitures scolaires. Dans un avis de mai 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'environnement et du travail. Lanxess a alerté sur la présence de substances dangereuses dans les fournitures scolaires et le bureau est recommandé d'étendre aux fournitures scolaires, la réglementation européenne relative à la sécurité des jouets. Au mois de septembre, ce risque était confirmée par les résultats d'une étude publiée par l'association de consommateurs, UFC, que choisir. Il y a 6 ans, cette association avait déjà alerté les pouvoirs publics, aucune mesure n'avait alors été prise. Au mois de décembre dernier vous avez répondu à mon collègue Pascal Alizart qu'il existait déjà une réglementation européenne suffisante je substances chimiques et annoncé une enquête de la DGCCRF. S'agit tout de même de conservateur allergisant de perturbateurs endocriniens de substances cancérigènes. Aussi, j'aurais souhaité savoir plus précisément les moyens dont dispose la DGCCRF pour contrôler les fournitures scolaires et permettent qu'à la rentrée prochaine, les familles et l'assurance que les fournitures ne contiendront plus le produit dangereux. Quel que soit leur provenance géographique. Je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Laurent. Roland Lescure Ministre délégué chargé de l'industrie. Si madame la présidente, monsieur le président. Babary merci pour votre question. Le marché français des fournitures scolaires coup une vaste gamme de catégorie de et de produits. Certaines d'entre elles peuvent être considérés comme des jouets et relève donc de la directive européenne relative à la sécurité des jouets mais la plupart d'entre elles ne sont pas des jouets. Compte tenu de leur absence de valeur ludique aussi n'est pas possible d'étendre à toutes les fournitures scolaires les dispositions réglementaires exit exigible pardon pour les jouets. Pour autant, la sécurité des fournitures scolaires et je pense que vous l'avez dit, à défaut de texte spécifique est assuré au travers de l'obligation générale de sécurité définies par une directive sur la sécurité générale des produits qui a été transposée en droit national dans le compte de la consommation. Par ailleurs, les matériaux et substances chimiques qu'elles contiennent sont encadrés réglementairement par un règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation. Les restrictions de substances chimiques règlement dite riche. Et un règlement relatif à la classification et d'étiquetage à l'emballage des substances et des mélanges. CLP textes prévoient respectivement des restrictions d'usage pour les substances les plus dangereuses, ainsi que des mentions obligatoires d'étiquetage, le cas échéant. Le gouvernement qui est très attentif à la protection des consommateurs et notamment des plus jeunes d'entre eux. Notamment pour ses produits qui concernent, par nature, un public vulnérable a pris note avec la plus grande attention de la vie de l'c'est ce que vous avez mentionnées relatif à l'expertise. Or, évaluation des risques relatives à l'état de connaissance sur la présence ou l'émission de substances dangereuses dans les fournitures scolaires et de bureaux à leur impact éventuel sur la santé, la DGCCRF, je vous le confirme renforcera le contrôle de ces produits et, dès cette année via une enquête dédié une synthèse de cette enquête sera ensuite transmise à l'. Afin que cette dernière dispose de données supplémentaires pour évaluer les risques sanitaires en cause. Merci beaucoup monsieur le président, ma Paris vous avez 45 secondes. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre. Le souci que que j'avais en, en posant cette question, c'est évidemment la rentrée prochaine. Je n'ignore pas la demande fait à la DGCCRF. Il se trouve que j'ai interrogé. Les personnels de la DGCCRF. Le problème c'est celui des moyens. Vous le savez bien, pour cette. Pour pour pour ses équipes, mais aussi la difficulté qu'il y a à faire les contrôles, faire une analyse faire des rapports, c'est bien faire les contrôles sur la masse de produits qui viennent. De l'extérieur c'est évidemment compliqué, mais on ne peut pas imaginer qu'à la rentrée prochaine. Les familles. Découvrent encore dans la presse des études qui font apparaître la présence des substances dangereuses, dont j'ai parlé. Jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Qui serait préjudiciable aux enfants. Merci. Merci la parole est à madame Elsa Schalke. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur un sujet majeur pour les finances de nos collectivités territoriales, l'exclusion des dépenses. D'acquisition d'aménagement et d'agencement de terrain dans l'assiette du FCTVA depuis le 1er janvier 2021. Ce sujet, nous l'avons évoqué ici à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle, nous avons voté la réintégration de ces dépenses pour les communes et leurs groupements à 2 reprises en juillet lors du PLFR mais également en décembre au moment du budget lors des débats budgétaires. C'est le ministre des Comptes publics qui reconnaissaient qu'il était nécessaire de revoir la situation malheureusement dans le cas du 49 3, le gouvernement n'a pas retenu l'amendement du Sénat qui reprenait pourtant les attentes et les besoins des collectivités territoriales, des associations d'élus d'élus locaux ainsi que les engagements gouvernementaux. Aussi je voudrais à nouveau ce matin me faire l'écho de cette attente forte de la nécessaire révision de l'assiette du FCTVA, on le sait cette exclusion porte préjudice à l'investissement local alors même que nous savons que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public, comme vous le savez Monsieur le Ministre, les conséquences financières pour les communes sont lourdes et ceci se rajoute un contexte financier particulièrement compliquée pour les communes qui sont touchés par l'inflation et par l'augmentation considérable du coût de l'énergie. Monsieur le ministre, il est impératif de mettre fin au discours contradictoires, d'un côté, encourager l'investissement local et demander aux communes de réaliser des travaux. Pour agir et pour agir, notamment pour la biodiversité et de l'autre, de modifier les règles de financement et il est impératif que le principe d'autonomie financière des collectivités retrouve une réalité dans notre pays, d'où ma question qui est très simple quand réintégrer vous ces dépenses d'aménagement et d'agencement de terrain au sein du FCTVA je vous remercie. Merci madame la présidente, madame a la sénatrice chaque pas de contradiction, mais la réalité au jour le jour de l'action publique qui vise oui certes à promouvoir l'investissement mais en préservant évidemment les équilibres budgétaires de la nation et l'efficacité d'une mesure, vous le savez, de de de fin 2020 puisqu'elle avait été votée dans le cas du projet de loi de finances pour 2021 qui vise à automatiser la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette automatisation pardon a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissements éligibles et certains comptes qui enregistre des dépenses auparavant éligibles n'ont pas été retenus. C'est notamment le cas du compte 212 agencement et aménagement de terrain dans la mesure où il comporte des dépenses hors taxes qui sont elles-mêmes inéligible au FCTVA Taylor, vous l'avez dit, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont pas éligible certaines dépenses pour autant réalisés par les collectivités dans le cadre du projet d'aménagement sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds, c'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbain. Qu'ils soient fixés au sol ou non des paires de buts filets de tennis panneaux d'information et qui, quant à eux, relèvent du compte 21 88 autres immobilisations corporelles les dépenses qui relèvent d'une imputation compte 21 58 Ostrava nation matériel et outillage technique comme les dépenses relatives à l'achat d'un tracteur ou encore les travaux d'éclairage du stade municipal, sont elles aussi éligibles au FCTVA. Par ailleurs, vous le savez les dépenses relatives à la voirie sont également éligibles. Si le principe d'inclure des dépenses des comptes 211 terrains et 212 agencement et aménagement de terrains. Vous l'avez dit, avait fait l'objet d'amendements. D'amendements pardon et d'échanges pendant les débats du PLF pour 2023. Ces mesures avaient été écartée au regard de leurs conséquences budgétaires avec un surcoût estimé à plus de 500 millions d'euros. Allons à l'encontre du principe de neutralité budgétaire de la réforme considérée dans sa globalité. Cette réforme s'avère favorable à l'investissement public local pour la bonne mise en oeuvre de la réforme de l'automatisation. Une évaluation de ce coup de ce dispositif est en cours de réalisation par les services de la direction générale des collectivités locales pardon et de la direction générale des finances publiques ces éléments seront présentés au printemps 2023. Merci, monsieur le Ministre. La parole est à monsieur Éric Bocquet en remplacement de sa collègue Michelle Gréaume. C'est bien cela. Merci présidente. Monsieur le Ministre. Mes chers collègues. Depuis plusieurs mois nos compatriotes salariés des services publics belges nous alerte sur les conséquences d'une modification à venir de leur statut fiscal. De quoi s'agit-il. Actuellement, une personne de nationalité française résidant en France et travaillant dans les services publics non concurrentielle belge est imposable en France. Or, une nouvelle convention de l'objectif est d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Signé, entre nos deux pays revient sur cette disposition à son application puisqu'elle n'a pas encore été ratifié ses salariés et nous parlons là de plusieurs milliers de personnes devront payer leurs impôts en Belgique. Ceci est lourde de conséquences pour des femmes et des hommes employer des hôpitaux, des écoles les structures médico-sociales et qui verront leurs revenus baisser de 25 à 30% les impôts sur le revenu en Belgique étant nettement supérieur au nôtre. au nôtre. Ce sont des projets de vie à long terme qui sont remises en cause. Nombre d'entre eux ont souscrit des prêts immobiliers par exemple sur la base de revenus et de capacité d'emprunt risquant d'être subitement d'évaluer et s'inquiètent à juste titre pour leur avenir. Une solution existe toutefois qui a déjà été mise en oeuvre en 2012 lors de la suppression du statut fiscal frontaliers contraint de payer leurs impôts en Belgique les travailleurs français du secteur privé belge déjà sous statut frontaliers ont bénéficié d'un délai leur permettant de continuer à payer leurs impôts en France jusqu'en 2033. À l'époque la modification du statut fiscal n'a été immédiatement appliquée qu'aux nouveaux frontaliers. Les employés français du secteur public belge qui ne remettent pas en cause la modification de leur statut fiscal souhaitent tout simplement bénéficier du même délai et des mêmes dispositions afin d'anticiper la baisse de revenus à venir. Aucune réponse précise ne leur encore été apportée, mise à part l'annonce d'une hypothétique et lointaine modification de la législation fiscale belge non confirmées, de l'autre côté de la frontière et semble-t-il une nouvelle fois repoussée cette vague promesse ne peut lever les craintes bien légitimes. Ma question est donc simple et précise, monsieur le ministre et j'espère que votre réponse le sera tout autant. Comptez-vous accéder à la demande des salariés français concernés de bénéficier des mêmes délais et dispositions que leurs collègues du privé en 2012. il y a quelques semaines dans cet hémicycle avec votre collègue, votre collègue pardon le sénateur Jean-Pierre Decool. Comme vous le savez, vous l'avez dit, la France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021, une nouvelle convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Destinée à remplacer celle en vigueur depuis 1964. Elle préserve le régime spécifique des frontaliers prévu au protocole additionnel à l'actuelle convention. Comme toute conventions fiscales bilatérales. Elle sera soumise au Parlement pour ratification. S'agissant des rémunérations de sources publiques. La convention franco-belge repose sauf exceptions sur le principe de l'imposition par l'État qui verse ses revenus. Ceci explique que la nouvelle convention prévoit que les salaires des personnes travaillant en Belgique pour une entité publique belge soit taxé en Belgique même si elles habitent en France. La reine inverse évidemment sera également vrai ne pourra que rendre plus attractif l'emploi public. De notre côté de la frontière dans des secteurs comme la santé et l'éducation qui sont décisifs pour le développement des zones frontalières. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une règle de bon sens qui évite qu'un État ne subventionne indirectement l'autre État pour payer à sa place. Des fonctionnaires qui seraient recrutés. De l'autre côté de la frontière. Je comprends que vous partagez ce constat, même si vous l'avez dit pour les résidents de France. Seule une catégorie des travailleurs verra son régime d'imposition modifié par les futures dispositions conventionnelles. Il s'agit des résidents français possédant la seule nationalité française percevant des traitements public de source belge exerçant leur activité en Belgique. Ses revenus sont imposables en France et seront imposables en Belgique par l'application de la nouvelle convention afin d'atténuer les effets de ce changement vous suggérer que l'Arago nouvelle ne s'appliquent qu'aux nouveaux travailleurs. Malheureusement cette comparaison a ses limites quand vous la comparer à celle dite des frontaliers depuis 2000. Tout d'abord, il s'agissait d'un régime historique. Qui visait à traiter la situation particulière. Des personnes en activité professionnelle requiert de franchir régulièrement la frontière ce régime contraint la France à verser une compensation financière. Le régime. Par ailleurs le régime et enfin le régime des frontaliers a vocation à disparaître, y compris pour les personnes qui étaient éligibles en 2011, ce sera le cas à partir de 2034. Monsieur, Monsieur le Ministre, j'ai quand même vous donner un bon point pour la gestion du temps, ne vous inquiétez pas. Oui oui vous avez rattraper complètement. Et puis je vous avez mis la pression alors donc. La parole est à madame Martine Filleul. Merci madame la présidente, madame la ministre, dans une tribune parue en décembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale. L'état dramatique de l'école et la comparer un Champ de ruines. La publication de l'indice de position sociale permet maintenant avec force information de partager ce constat alarmant. Oui, le principe d'égalité et très largement défaillant le déterminisme social frappe dès le plus jeune âge. Sont toute perspective d'égalité des chances et au sommet d'une hiérarchie scolaire qui ne dit pas son nom trône l'enseignement privé et l'enseignement catholique dans le département du Nord avec un IPS de 97 soit 6 points de moins que le niveau médian au niveau national, les voyants sont au rouge. À Lille, où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les voyants sont au rouge, très vif, puisque la moitié des établissements y'affichent un IPS inférieur ou égal à 93 avec des différences très importantes entre école et quartiers Madame la Ministre. La question n'est pas simple. Contrairement à l'habitude. Dites-moi quelles réformes structurelles porte ce gouvernement pour rétablir l'égalité républicaine et la mixité sociale dans nos écoles en combattant effectivement la ségrégation qui est à l'oeuvre. Merci la parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Bonjour, madame la Ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs. Les sénateurs, madame la sénatrice Martine Filleul, vous avez raison, la seule manière de. Lutter contre les inégalités compte les déterminismes sociaux c'est de s'attaquer à la mixité sociale à l'école et c'est la mère des batailles et vous avez également raison madame la sénatrice. Ce n'est pas un exercice aisé et la première des étapes c'est évidemment la transparence, la connaissance de ces IPS les rendre publics bien sûr mais ça ne suffit pas que de savoir maintenant il faut voir comment on Nièvre. Temps court moyen temps long mais comment Nièvre et pour ça, madame la mini-, je peux vous assurer que le ministre de l'Éducation nationale en a fait un combat, un combat sincère, puisque la stratégie mise en oeuvre, elle doit d'abord être construite sur nos territoires puisque les différences sont criantes, mais elles sont très inégale d'abord avec les avec les maires, avec les présidents de départements en réalité avec les associations de parents d'élèves, les parlementaires et tout ça se déclinera avec des mesures fortes au sein d'établissements scolaires. La première politique mise en oeuvre pour aller chercher une justice sociale plus forte, une mixité sociale plus forte au sein des au sein des des territoires a été expérimenté entre autres dans l'académie de Lille. D'abord la révision de la carte de sectorisation, on sait que c'est pas un exercice facile mais pour autant nécessaire et ambitieux qui s'opère progressivement lorsque la géographie du territoire le permet, en s'appuyant sur des dispositifs de secteur je pense évidemment aux multi-collèges au multi-lycée ou encore au jumelage d'établissements la transformation effective des conditions d'affectation et et l'accueil d'élèves boursiers dans tous les établissements. Des contrats de mixité avec lesquels les établissements scolaires s'engage à accompagner les élèves les plus fragiles socialement en mobilisant les cordées de la réussite ou encore le soutien du tutorat du mentorat les stages de réussite l'enrichissement de l'offre pédagogique et l'implantation de cursus d'excellence mais nous savons madame la sénatrice. Que tout cela ce sont des des des éléments complémentaires des dispositifs qui corrigent mais dans le fond la plus forte et la réponse. La plus nécessaire, c'est évidemment le développement de la coopération avec les collectivités territoriales pour une prise en charge des transports scolaires, c'est la mobilité aussi qui freine les frais d'hébergement ou de restauration afin de faciliter une mobilité plus forte des élèves et favoriser la mobilité sur l'ensemble du territoire. La mobilisation des acteurs et nécessaire. je vais me tenir évidemment et ce sera que la première je je ferais l'effort nécessaire. Madame la présidente. Allez-y, allez le débat sera organisé le 1er mars, madame la sénatrice à votre initiative de mémoire et le le ministre aura l'occasion de rentrer plus en détail sur ce plan. Merci. Même si elle vous avez 36 secondes. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il faut une réforme structurelle et globale, ambitieuse pour faire évoluer notre système éducatif et pour endiguer cette ségrégation, je me permets d'insister sur la question de la carte scolaire, il faut la transformer en profondeur. Cesser la fermeture systématique, auquel nous assistons de classe et faire preuve de plus d'exigence de fermeté par rapport à l'enseignement privé, donner des moyens aux zones d'éducation prioritaire et mieux rémunérer les enseignants. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Marie Mercier. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais vous parler du harcèlement scolaire à peu près on pense un million de jeunes seraient victimes de ce cauchemar à la fois à l'école bien sûr, mais aussi en dehors, à cause des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Ces enfants vivent un véritable calvaire qui mêle à la fois la violence la répétitivité mais surtout l'isolement. Qu'est-ce qu'ils disent. Personne ne m'écoute. Personne ne me croit alors je vais m'appuyer sur le cas d'un jeune de mon département que nous appellerons Maëlle. Ses parents ou des, j'ai beaucoup de mal à faire admettre qu'il y avait harcèlement scolaire et maintenant il faut qu'ils se battent contre les institutions. Pourquoi, parce que c'est le jeune enfant harceleurs qui a lui aussi probablement besoin d'aide mais qui va rester dans l'école et c'est Maëlle qui est contraint de quitter son école aussi Madame la Ministre je voudrais vraiment savoir quel est votre ressenti sur cette question qui gâche la vie de tant de nos enfants qui leur fait vivre un vrai enfer, alors ne me parlez pas des dispositions phares les axes, les mesures, les piliers, tout ça on connaît, qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire pour aider et sauver nos petits-enfants. Merci, cher collègue, la parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs Madame la sénatrice. Vous avez raison, je ne veux pas vous parler ni de fard ni de la loi Balanant de ni des programmes de lutte, même s'ils sont nécessaires parce que c'est une première réponse et on sait à quel point aujourd'hui pour que les parents pour que Mel puissent avoir une écoute. Accompagnée, il faut former évidemment les encadrants et mobiliser l'ensemble des maillons de la chaîne éducative. Les enseignants, les CPE, les infirmiers, les infirmières scolaires et évidemment tous ceux qui encadrent au quotidien nos enfants mais madame la sénatrice, le harcèlement est un fléau. C'est un fléau qui tue c'est un fléau qui tue qui brise des familles pour 2 raisons, la première c'est qu'il ne s'arrête jamais. Ce qui vous prend aux tripes, il vous il rentre dans votre tête et finalement il vous Brice et dur de se rendent compte que finalement la honte doit s'inverser. C'est dur de dire à un jeune adolescent qu'il n'y est pour rien. Et pour cela, hein vous m'avez demandé mon intime conviction mon intime conviction c'est que ce jeune Maëlle n'a pas à partir de son établissement. En réalité, un jeune doit être accompagnée. Il est la victime et la victime n'a pas à partir, si ce n'est malheureusement le risque de prendre de vivres. L'impression d'être deux fois pénalisé ou en tout cas deux fois puni alors que ce n'est pas le cas. Madame la sénatrice. Je crois que c'est un fléau de notre temps. Il est renforcé par une. Une société qui est aussi parfois plus violente avec ses réseaux sociaux puisqu'il n'y a plus de frontières que ce qui se passe. En ligne se retrouvent dans les cours dans les cours d'école. Ce qui se retrouvent dans les cours d'école se retrouvent dans sa chambre le soir tard, sans ses parents malheureusement parfois des parents démunis qui n'ont même pas conscience de ce que vit leur fils ou leur fille et donc si j'avais. À pour le coup bien sont trop petits. Mais si j'avais peut être une un message une force ne jamais avoir peur ne jamais avoir honte le dire et quand on est quand on est le la le camarade quand on est parfois l'adultes encadrants hé bien parler vaut mieux mobiliser plus de monde que pas assez. À chaque fois que nécessaire et surtout se doter d'une grande prise de conscience sociale puisque ça tue nos enfants aujourd'hui.

le fait que Maelle n'a pas à changer d'école, c'est bien ce que vous avez dit donc Maëlle doit rester dans son école. Vous avez parlé aussi de l'ensemble des maillons de la chaîne et là je voudrais vous faire une suggestion. Il y a des comités d'éducation dans les collèges, dans les écoles mais très souvent, le maire n'est pas impliqué puisque l'école est fermée, quand c'est pas l'école qui est fermée, c'est le collège et vice-versa. Il faut faire rentrer les maires puisque les maires sont les employeurs, des Atsem les maires assure la cantine, il s'occupe de 30 du transport scolaire et c'est là aussi que l'enfant souffre donc je compte sur vous pour que les écoles s'ouvre et compte la psychologue viennent au moins le maire soit invité à la réunion. Merci madame. Merci. La parole est à madame Angèle Préville. Merci madame la présidente, madame la ministre. Alertés par des élus du département du Lot, je souhaite vous interroger sur le financement de la pédagogie dans nos collèges. Depuis plusieurs années, l'État semble se désengager, laissant les collectivités territoriales assumer toujours plus de dépenses qui normalement lui incombe. Le financement des actions pédagogiques ne relève pas de la compétence des collectivités locales bien sûr. Il semble par ailleurs qu'aucune logique nationale ne prévalent sur le financement de ce volet pédagogique plus généralement d'une année sur l'autre, d'une académie à l'autre, d'une collectivité territoriale à une autre, les règles du financement de la pédagogie sont devenus très variable. La dotation des départements et destiné à la construction et à l'entretien des collèges mais le département du Lot subventionne également des projets éducatifs sportifs, culturels et de prévention. Pour l'instant, le département du Lot augmente ses subventions au profit des pros des des projets pédagogiques, voire même au financement de la pédagogie elles-mêmes à savoir l'achat de manuels scolaires si cela résulte d'un choix politique engagée supportable. Jusqu'à présent il ne s'inscrira peut être pas dans la durée au vu du contexte économique difficile. Pourtant, les équipes éducatives devrait pouvoir compter sur des Budgets pérennes pour pouvoir construire sereinement des projets ambitieux pour les enfants ne de notre département. Monsieur Madame la Ministre n'est-ce pas à l'éducation nationale de donner aux établissements les moyens d'acheter les manuels les livres dans les CDI et de financer les sorties scolaires, autrement dit de financer la pédagogie, je vous remercie. Si la parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Préville. La question budgétaire. Et est souvent posée quand on parle d'école et vous avez raison. Aujourd'hui l'éducation nationale le océan c'est un, c'est le plus grand budget de l'État en 59 milliards d'euros, augmentation nécessaire. Et pas loin d'être inutile de plus de 6 pour 106% cette année mais il y a une répartition des compétences, qui est très clair. La responsabilité qui incombe et qui est fixé d'ailleurs par le code de l'éducation, mais la question, la question qui incombe aux communes aujourd'hui ou au bloc communal, c'est évidemment les locaux. Ensuite, on a l'État qui prend sa charge et ça part avec la rémunération des enseignants. Mais au-delà de ça, les crédits pédagogiques qui permet de financer les actions pédagogiques du 1er degré dans le cadre. Notamment de l'école. Il recouvre quand même madame la sénatrice, peut être l'idée qu'il y a un parcours de citoyenneté qui peut s'envisager aujourd'hui nous voyons un certain nombre de collectivités, d'ailleurs je les salue qui. Soutiennent des projets pédagogiques complémentaires, je pense aux classes découverte je pense à l'école hors les murs. Je pense aussi parfois parfois certains forums associatifs qui ont lieu dans, dans nos communes. Ce sont effectivement des désengagements des projets d'établissements qui sont soutenus par les élus locaux, parce que ce sont les premiers pour moi ce sont les les premiers bâtisseurs de cette citoyenneté. On a deux manières de voir l'école, l'école avec un grand E, soit c'est un lieu d'instruction exclusivement et donc la formation se fait exclusivement sur les fondamentaux pédagogique ça nous considérons que c'est un lieu d'éducation et donc d'éducation également à la citoyenneté. Au civisme et à l'engagement. Et à ce moment-là, effectivement, les projets soutenus par l'ensemble des élus, qu'ils soient d'ailleurs du bloc communal du bloc départemental sont des bien fait le point d'alerte et là je vais vous rejoins madame la sénatrice, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité qui n'est pas d'inégalité, en fonction des territoires et en fonction du coût des sensibilités politiques et vous voyez très bien à quoi je fais référence pour qu'il n'ait pas d'inégalité. Le président de la République a souhaité que ces projets d'établissements, soit plus nourris plus fort et donc a mis en place un fonds d'investissement pédagogique de 500 millions d'euros sur le quinquennat. Suite au CNR, je vous remercie. Merci madame Préville vous avez 26 secondes. Merci madame la présidente, mesdames Namyst Ministre merci pour votre réponse. Alors bien évidemment les collectivités comme les départements. Financent des projets pédagogiques complémentaires. Et j'espère que sur le fond dont vous nous avez parlé pourra servir à l'achat. De matériels pédagogiques proprement dit, quand on parle de manuels scolaires. C'est le cas et c'est vrai que on peut enfin j'espère que dans l'avenir. Les départements n'auront pas abonder ce qui est de la pédagogie elles-mêmes je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Daniel guéri. Madame la présidente, madame la ministre je souhaite attirer l'attention de monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse sur ses services départementaux qui étudie actuellement la carte scolaire pour 2023 2024. Un certain nombre d'élus sur notre territoire et destinataire d'un courrier, précisant que l'évolution des effectifs prévus à la rentrée prochaine pourrait rendre nécessaire un retrait de moyens dans une école. Il s'agit d'une approche purement comptable en aucun cas humain et tout le monde en est bien conscient. Et cela suscite l'inquiétude des élus et des parents d'élèves qui engage les actions au travers de manifestations, pétitions, point presse. C'est le cas dans plusieurs villes de mon département, l'Eure-et-Loir. Je souhaite par conséquent interrogé le ministre sur les conséquences de ces décisions qui s'imposent aux enseignants et aux élèves en unité localisée pour l'inclusion scolaire dites Ulysse et en particulier sur l'innocuité de traitement des enfants en situation de handicap dès lors qu'ils habitent en milieu urbain ou en secteur rural, les moyens mis à disposition d'un établissement sont totalement différents, selon qu'il se trouve dans une ville ou dans un village, ce qui est particulièrement vous en conviendrez choquant lors de la prise de ces décisions, cette administration sous-estime le fait que la fermeture d'une classe a pour conséquence d'augmenter le nombre d'élèves Ulysse dans les classes restantes compliquant voire décourageant. La tâche des enseignants très très investi, qui sont sans moyens pour accompagner ses enfants supplémentaires aussi à l'heure où la politique du gouvernement et de promouvoir l'inclusion en milieu scolaire, je souhaite connaître Madame la Ministre, les mesures concrètes mises en oeuvre, en particulier en milieu rural pour donner à tous ces enfants en difficulté les mêmes chances d'apprentissage et à tous nos enseignants la pluie nécessaire au bon exercice de leur mission. Merci la parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. beaucoup madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Vous savez comme vous sur mon territoire. À chaque fois que la question d'une fermeture de classe se pose évidemment, il y a les parents d'élèves qui se mobilisent souvent les équipes pédagogiques aussi parce qu'il voit les conséquences objectives d'ailleurs d'une d'une réorganisation de ce type-là. Et souvent, hé bien on s'y intéresse et ça crée de de de l'émotion est légitime, mais s'il y a un endroit où il n'y a pas à avoir d'analyse comptable. Je crois que c'est à l'école et au sein de l'Éducation nationale puisque je sais qu'on ne sait pas le comté sont. Quelle est la prévention qu'elle est le fruit je sais qu'on sait pas le comté. Je sais qu'on ne sait pas dire combien finalement ça évite de dépenses demain mais s'il y a un rêve français, c'est peut-être celui-là, celui du mérite de l'élévation par l'effort et celui de l'égalité devant l'accès. À la formation et l'éducation. Et c'est pour ça que 0 logique comptable, en tout cas pas au sein de l'Éducation nationale. Et malgré la baisse démographique et la singularité de nos nos territoires. Il est nécessaire aujourd'hui de continuer à accompagner chacun des des enfants quel que soit, c'est leur difficultés, vous parliez des classes Ulis en particulier. Aucune ne sera fermé l'année prochaine

11 postes en moins et effectivement là je parle de en moins. Et pour autant, la moyenne par classe le du taux d'encadrement et meilleur en Eure-et-Loir que dans la moyenne nationale. Mais ça ne veut pas dire que que il faut s'arrêter sur ces moyennes et sinon ça viendrait totalement contredire mes propos initiaux. C'est la question de l'ACF spécificités territoriales qu'il faut aller accompagner et donc pour revenir sur ces que la Suisse qui demande une attention particulière. Il est plus que nécessaire de regarder la les caractéristiques de la population scolaire mais aussi la mobilisation des et des élus locaux, elle est absolument essentiel. On sait que je veux dire la chaîne éducative et pédagogique dépend aussi de la mobilisation et la sensibilité de ceux-là. La question aussi de la distance. On sait que les questions de mobilité. Elles ont des conséquences sur, sur les enfants. La question de l'enclavement. La formation professionnelle sur le bassin pour voir les les continuités et effectivement peut être une spécificité qui est l'offre sociale. Et donc le travail avec l'ARS et les familles. Monsieur le sénateur. S'il n'y a une seule éducation à tenir si un seul investissement à faire, c'est celui de l'école en 1er lieu je vous remercie. Merci la parole est à madame Céline brûlant. Merci madame la présidente, madame la Ministre, la soustraction serait-elle l'opération préféré dans l'éducation nationale, 25% des postes supprimés nationalement dans les lycées le serait en Normandie qui perdraient 306 heures de dag dont 134 rien que pour la Seine Maritime. Le lycée Maupassant à Fécamp perdrait ainsi 98 heures pour 34 élèves de moins qu'à la dernière rentrée. Et dans cette équation aucun poste pour le retour des mathématiques annoncé pour tous les lycéens de première. Dans les collèges soustraction toujours avec fermeture de classe et effectif sur sa surchargé comme à Picasso à Harfleur ou Monet à gruger le Valace quant aux enseignants de technologie ils ont appris par les médias, la suppression de leur matière en sixième au motif de créer une heure de renforcement en français et en mathématiques dont que personne ne sait aujourd'hui qu'il assurera. Pour le primaire, 111 fermetures sont prévues en Seine-Maritime pour 79. Ouverture et les regroupements et les fermetures de classes en milieu rural se développe. Or nos villages aussi sont des zones prioritaires. L'argument démographique a bon dos. Surtout que le manque de remplaçants y compris pour des absences prévues accroît encore les effectifs dans les classes. Déjà 46 jours non remplacés depuis septembre à l'école. Thomas Pesquet du Fontenay.

mais nos enfants ont besoin d'enseignants, enfin comment faire de l'école inclusive une priorité avec la suppression de 4 postes d'enseignants dans les centres médicaux psycho-pédagogiques du Havre de Rouen ou de Dieppe ou avec des élèves relevant du Lys, ne pouvant plus être accueillis en 4ème au collège Victor Hugo en scène l'insuffisance des crédits sur lesquels nous avions alerté se confirme, Madame la Ministre cela conduit à mettre tous les besoins en concurrence dans une gouvernance de la pénurie alors que le seul objectif devrait être la réussite des élèves. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers collègues, je suis aussi très attachée au lycée de Fécamp. Je vous le dis madame la ministre, je vais vous donner la parole. La parole est donc à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Si beaucoup madame la présidente. Maintenant, madame la présidente. J'ai en plus la pression sur la réponse le le l'établissement de Pékin, mesdames, messieurs. Mais le coeur brisé, et le message. Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice brûlant. Vous parliez de soustraction. Il se trouve que c'est pas ma force les mathématiques si même si ce n'est l'élan cependant il y a une soustraction effectivement que vous avez, vous avez cité rapidement, c'est celle de la démographie, c'est pas une histoire de Bondo ou pas sur d'ici la fin du quinquennat, on aura 500.000 un demi million d'élèves en moins dans notre système scolaire. Effectivement ça appelle à des organisations à des évolutions mais là où je suis d'accord avec vous Madame la sénatrice. Il faut regarder ça avec l'une territorialité avec des besoins spécifiques en fonction des territoires et il n'y a pas de raison que les territoires ruraux soit plus impactées que des territoires plus dense où plus urbain cependant s'puisque la question se pose sur l'académie de Normandie, plus, plus particulièrement, il y a 5296 élèves en moins sur la rentrée 2023 plus concrètement sur la Seine Maritime. Depuis 2016, la baisse des des effectifs a été de 6747 élèves au 1er degré, passant de de 115.250 à plus de 108.447. Avec pourtant 270 postes qui ont été gagnées à la rentrée 2023, le, le département devrait perdre plus de 1000 élèves. Mais malgré ces baisses significatives, ce que je disais que j'étais pas, c'était pas mon fort. Et puis en fait c'est pas ce qui fait qu'on s'engage politiquement les mathématiques. Très sincèrement, peut-être pour d'autres, mais en tout cas moi c'est pas ce qui fait que je m'engage, ce qui fait que je m'engage, c'est la vision et l'importance de l'école, est ce que ça apporte en réalité dans la vie de jeunes qui parfois n'ont pas les mêmes chances du fait de leur famille, du fait du capital social de leur famille et du fait de leur territoire et moi ce que je vois c'est qu'il y a un taux d'encadrement qui quand même s'améliorent. Ce n'est pas parfait. C'est vrai mais on passe. On passe de plus en plus dans les zones. Hors zone prioritaire à un taux d'encadrement plus bas et s'agissant tout particulièrement du du regroupement pédagogique intercommunal de la fin de la forêt de donc le Hongrois Melville 1000 Bosc guerre ville il s'agit donc d'un RPI de 5 classes réparties sur 4 sites pour lesquels 88 élèves sont attendus à la rentrée 2022, les effectifs moyens de la classe et de 22 après la fermeture d'une classe les projections prévoient 70 élèves maximum d'ici 2 ans. Et quant à la situation de l'école Tome Thomas Pesquet madame la présidente et Madame la sénatrice. Vous avez parlé effectivement d'une situation plus tendue plus grave. Il se trouve que la situation est en train de s'apaiser depuis 3 semaines. Puisque l'installation durable d'une remplaçante. Et est arrivée et elle elle sera assurée jusqu'après le retour des vacances d'hiver pour madame la sénatrice. Nous avons besoin d'enseignants, d'hommes et de femmes devant les élèves et c'est clair que. Aucun outil numérique aucun outil pédagogique ne remplacera ça et pour le coup vous avez la. Vous avez ma conviction que le ministre de l'Éducation nationale se bat et je pèse mes mots, pour aller recréer de la la d'évocation accompagner ces vocations et cette attractivité puisque c'est la condition de la réussite. Je vous remercie.

merci madame la présidente, madame la ministre je souhaite attirer votre attention sur la situation préoccupante du lycée d'Darchy cours d'Hénin-Beaumont pour la prochaine rentrée scolaire, les professeurs de ce lycée ont toujours eu à coeur de mettre en application les principes de leur projet établissement intitulé Culture ambitions ambitions réussites. L'action de la communauté éducative du lycée d'Achicourt et guidée par les principes des valeurs de la République et par la volonté de faire réussir les élèves. Cette action passe par la richesse d'offres de matière de de spécialité d'options culturel, artistique, linguistique et sportive de projets comme les échanges internationaux des projets de

pour la classe de seconde. La Russie des plus fragiles des élèves peut de ce fait être malheureusement compromise après cette forte mobilisation de la communauté éducative, les options qui font la richesse de l'établissement sont finalement maintenu mais avec une quantité horaires diminués et certaines options sont voués à disparaître en 24 et 25. Comment lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la discrimination aux origines quand on réduit ainsi drastiquement les moyens les plus efficaces de cette même lutte dans un bassin, fortement marquée par la désespérance sociale. L'an dernier déjà la mobilisation des personnels avait permis de récupérer des heures d'enseignement indument supprimer. Il est primordial d'augmenter les moyens dans l'académie de Lille qui connaît la plus grande réduction de moyens dans le second degré pour la 5ème année consécutive. Je vous demande Madame la Ministre de mettre les déclarations de monsieur Pap Ndiaye notre ministre en adéquation avec les actes police politique du gouvernement et ainsi de revenir sur la diminution des moyens octroyés à l'académie de Lille et en particulier au lycée d'Achicourt d'Hénin-Beaumont. Il en va de l'avenir de ses élèves. Bonjour, merci. Merci, cher collègue, la parole est à madame Sarah et la Yaris secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, je vais aller droit au but. Vous avez posé la question sur le lycée d'Achicourt et d'abord c'est un lycée qui a perdu un certain nombre d'élèves, on est passé de 1751 1659. C'est un établissement qui a perdu 5% de ses, de ses élèves en 2 ans alors que, au niveau national, le nombre de lycéens. A plutôt augmenté de 0,8% sur ces 2 mêmes années. Malgré ça les ajustements de la dotation de ce lycée s'inscrivent aussi dans ce contexte ce lycée effectivement il vous l'avez dit, vous l'avez souligné par la force de la mobilisation de son équipe pédagogique aussi à une palette très large de formation, notamment je pense en plus à la section européenne à la section binational. Aux différents BTS aux classes aux spécialités numérique et sciences. Et ce lycée, il a un nombre d'heures par élève. Qui. Est de 1,26. Il s'agit du taux le plus favorable de H nationale qui est que de 1,18. Au niveau du lycée en pré bac. Il est déjà plutôt bien accompagné madame la sénatrice et ces, ces 2 indicateurs montrent que, malgré ça, parce que tout à l'heure je disais que il ne faut pas avoir l'éducation nationale comme quelque chose de mathématiques mais il faut regarder les spécificités du territoire et des besoins. Les services académiques suivent la situation de ce lycée avec attention et prendront et j'en prends l'engagement prendront si besoin en compte des ajustements nécessaires à la rentrée 2023. En général c'est discuter mais vous le connaissez, vous savez très bien la procédure ou que là vous la maîtriser, madame la sénatrice en général en juin juillet au moment. Ah la, vers la fin de l'année, et plus généralement le taux d'encadrement sur l'académie de Lille c'est quand même un des plus favorables aujourd'hui qu'on est sur le niveau national. Alors il y y a 2 manières de voir, soit on tire tout le monde vers le haut, soit vous dire tout le monde vers le bas. Moi je suis plutôt de ce qui a envie de tirer plutôt tout le monde vers le haut. Alors au lieu de comparer, gardons les plus beaux projets sur nos territoires accompagnons-le avec beaucoup d'Intelligence et voyons comment on peut sécuriser c'est joli, c'est joli climat aussi Serge July climat scolaire en tout cas dans cet établissement parce que du coup j'ai regardé dans le détail et faisons que avec les services académiques, on trouve les réponses nécessaires. Je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Thani Mohamed Soilihi. Merci madame la présidente. Madame la ministre je souhaite attirer votre attention sur la situation très critique. Que rencontre l'association transition pro de Mayotte. Vous le savez, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé les commissions paritaires interprofessionnelles régionales dénommée Association transition pro qui se sont substitués aux fonds de gestion de congé individuel de formation, il faut j'ai SIP. En 2020, cet outil qui permet la reconversion professionnelle des salariés du privé est très récent. À Mayotte, qui n'a connu ni congé individuel de formation ni foi je la quote-part de la dotation du, du projet de transition professionnelle alloués aux associations transition pro est calculé à partir de la masse salariale de chaque territoire. Or à Mayotte. Ces données ne sont ni stabiliser ni fiables aussi la dotation actuelle ne lui permet pas de réussir à répondre aux besoins d'un public croissant et l'a contraint un autre à sous-. Traiter une partie de ses dossiers à la Réunion. Cette sous-dotations met en péril l'existence même de la structure puisque, faute de moyens, l'association devra cesser toute activité en mars 2023, c'est-à-dire dans moins de un mois dans un contexte insulaire fortement marquée par des retards structurels de développement, notamment en matière d'emploi, de formation et de professionnalisation de la population active. Je vous demande Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement entend prendre pour sauvegarder l'existence de l'association transition pro de Mayotte. Merci, cher collègue, la parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup madame la présidente, monsieur le sénateur, messieurs les sénateurs. Je vais aller droit au but. Monsieur le sénateur, et je peux vous assurer que le gouvernement soir à vos côtés sans faille pour garantir le droit d'accès au dispositif de transition professionnelle, sur l'ensemble du sur l'ensemble du territoire mahorais et pour l'ensemble des salariés. Qui permettra le développement de l'île. Bien sûr, monsieur le sénateur, au-delà de notre mobilisation, je vais vous donner quelques éléments qui m'ont été portées par le ministre du Travail, compte tenu de la typologie de la question. Vos préoccupations sur transition prend de Mayotte sont aujourd'hui identifiés et suivis par les services du ministère et comme vous le rappelez, le système actuel de définition des frais de gestion des de des transitions pro prend effectivement difficile rend difficile le bon fonctionnement de cette structure. Mais monsieur le sénateur, les multiples alertes et sollicitations que vous avez pu nous faire part nous amène aujourd'hui à établir des évolutions nécessaires pour vous, pour accompagner d'abord la dotation qui a été votée par France compétences et versée aux transitions pro pour financer les projets répartis entre elles au prorata de la masse salariale par région des frais de gestion au pourcentage de la dotation reçu soit ensuite négocié entre transition pro et les services déconcentrés. Il s'avère que ce mode de calcul ne permet pas ah transition pro-Mayotte de bénéficier des frais de gestion suffisant pour assurer le paiement de locaux et de charges courantes et de 2 effectif qui permettrait à priori d'assurer les missions de transition pro dans ce qu'on cesse dans ce contexte, Monsieur le Sénateur. Une convention de partenariat signé entre transition pro-Mayotte et transition pro-réunion permet effectivement d'instruire les derniers dossiers de demandeurs. Prenant fin le 31 décembre 2022 son renouvellement a été demandée par la des est en cours d'instruction. Quant à la situation financière. Dans un premier temps une solution va être mis en oeuvre pour remédier aux difficultés immédiates. Monsieur le sénateur, mais il faut aussi penser à l'après et pour cela, la ministre déléguée Carole Granjean. Prendra en charge spécifiquement cette alerte, monsieur le sénateur et contact avec les services départementaux pour trouver une solution à long terme. Merci madame la ministre monsieur Mohamed Soilihi, vous avez 24 secondes. Oui merci ma Madame la Ministre pour. Ses, ses engagements. Vous savez notre ils rencontrent des difficultés, mais nous nous battons et les administrateurs de transition pro se battent et. Je vais avec plaisir le faire-part de cette de cette bonne nouvelle. la parole est à monsieur Cyrille va. C'est ça. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question était originellement adressé au ministre du Travail, à qui j'adresse mon plein et entier soutien enfin ses attitudes qui ne dort pas les politiques. Voilà elle porte en effet sur l'opportunité de créer un statut spécifique aux travailleurs saisonniers. Essentiel aux activités touristiques et participant à l'excellence de la France en matière et travailleurs saisonniers ont pour spécificité d'être plus réactif et d'exercer plusieurs métiers de manière intermittente. Ainsi, sur une année un saisonnier disposera typiquement de de contrats d'une durée moyenne de quatre mois avec des amplitudes horaires importantes et exposant souvent à des critères de pénibilité. Ces contrats sont habituellement séparées par des périodes d'inactivité d'environ 2 mois en inter-saison à la fois par nécessité de se reposer mais aussi faute de trouver un emploi durant ces périodes de baisse d'activité si leur employeur font des efforts pour favoriser les CDI. L'essence même du tourisme fait qu'ils restent rares. Cette situation entraîne alors des effets de bord impactant les saisonniers. C'est le cas en matière de recherche de logement ou encore avec la réforme de l'assurance chômage qui requiert désormais de cotiser durant 6 mois qu'on ne IV par le passé. De même, alors qu'auparavant seuls les périodes travaillées durant les 6 derniers mois été comptabilisés des périodes d'inactivité sont maintenant prises en compte pour établir une moyenne sur 10 mois. Les droits sont en outre ouvert sur 10 mois contre six avant la réforme. Si l'objectif était de lutter contres les personnes profitant du système, qui cherchait à travailler le moins possible ces nouvelles règles un de nombreux saisonniers qui sont simplement contraint par la saisonnalité de leur activité n'ont plus accès à l'assurance chômage ou tout du moins, reçoivent une allocation dont le montant est légèrement diminué. La réforme des retraites pourrait elle aussi les pénaliser. En effet, s'il est prévu d'instaurer une retraite minimale de 1200 euros. Cette mesure ne vaut que pour les carrières complètes. Or les saisonniers n'en ont que rarement du fait des périodes d'inactivité entre leur contrat. Il devrait donc travailler jusqu'à plus de 67 ans, alors même qu'ils exercent la plupart du temps des métiers physiques. De surcroît, s'il pouvait être attendu à un départ anticipé grâce à la pénibilité de certaines de certains métiers saisonniers, il semble que telle ne sera pas le cas puisque les seuils définis par la loi ne sont problème maman pas atteint, du fait de la permittence de leur activité. Aussi Madame la Ministre je souhaite savoir si le gouvernement envisage l'adaptation assez de réformes pour mieux prendre en compte les spécificités de contrat saisonnier. Faute d'adaptation, il est à craindre une désertification de ces métiers, ce qui entraînerait une dégradation de leur qualité du tourisme français qui est pourtant l'un des plus performants au monde. Plus largement, je m'interroge sur l'opportunité de créer un statut spécifique au métier saisonniers qui pourraient s'inspirer de celui des intermittents du spectacle. Je souhaiterais donc connaître la position du gouvernement à ce sujet, je vous remercie. Alors, chers collègues, je vais juste vous rappeler que ces deux minutes et pas 2 minutes 30. Vous imaginez si tout le monde avait fait ça à à quelle heure on termine, on doit terminer absolument 13h donc. Il faut voir avec vos collaborateurs pour si vous cible vos, vos questions, merci. La parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup madame la présidente, monsieur le le sénateur. Il se trouve qu'il y a un point commun entre la Haute-Savoie et la Loire-Atlantique c'est l'attractivité touristique pour l'une montagne pour l'autre littoral mais la question des saisonniers se pose et se pose pour plusieurs raisons aussi chez nos agriculteurs pour être. Très explicite et vous apporter la réponse du ministre du Travail, monsieur le sénateur, la réforme de l'allocation chômage. Ni à jouer en réalité que de façon marginale sur les emplois saisonniers. La réforme du calcul de l'allocation. On a commencé à s'appliquer qu'à partir du 1er octobre 2021. Quant au passage de 4 à 6 mois que dont dont vous parlez il peut avoir touché les saisonniers de carrière qui généralement travailler plus de 6 mois pendant l'année

la durée des contrats d'intérim et notamment à notamment augmenter significativement. Et le gouvernement s'inscrit tout à fait dans la démarche de soutien de la filière saisonnière, que vous appelez de vos voeux plusieurs mesures de soutien au secteur du tourisme en particulier ont été mis en place. en particulier aux échanges au sein du plan destination France que vous connaissez, monsieur le sénateur, et de nouveau guichet d'accueil. Et d'orientation des saisonniers qui ont été installés dans les zones les plus touristiques. Ce plan doit se poursuivre et couvrir l'ensemble des bassins et depuis octobre 2022, le pôle emploi a également mis en place un certain nombre d'agences de viviers de viviers de demandeurs motivé pour avec des compétences transversales pour accompagner aussi les métiers du. Du HCR donc hôtel hôtellerie. Commerce restauration et par ailleurs, le service public de l'emploi et les Opco ont commencé à nouer aussi un certain nombre de partenariats. Monsieur le sénateur, je ne sais pas si l'époque veut des régimes spécifiques. Mais ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui les métiers saisonniers, qu'il soit agricole ou touristique, appel des contraintes supplémentaires et un accompagnement particulier, que ce soit la question du logement. Quand vous avez un mois de votre salaire qui passe. En loyer ou encore la pénurie, fait que nous devons traiter cette question de manière systémique et le, je suis sûr que le mini sera à vos côtés pour travailler sur cette question plus en profondeur. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Alors je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h 30 pour l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. La séance est suspendue.